En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- huit voix pour, aucune voix contre, cinq bulletins blancs -à la reconduction de M. Jean-Bernard Lévy dans les fonctions de président-directeur général d'Électricité de France. L'ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe La République En Marche, de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi examinée aujourd'hui répond à un objectif dont on ne peut douter de l'intérêt, puisqu'il s'agit de faciliter les démarches des administrés et d'agir pour leur pouvoir d'achat. Cette possibilité est attendue par nos concitoyens, qui souhaitent obtenir davantage de souplesse et ainsi pouvoir résilier leur contrat de complémentaire santé sans frais et à tout moment au terme de la première année de souscription. Il s'agit de mesures à la fois pragmatiques et concrètes, qui s'inscrivent dans la continuité de la faculté, offerte aux assurés par la loi relative à la consommation de 2014, de résilier leur contrat d'assurance automobile ou emprunteur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription. Je ne puis que regretter le sort réservé à ce texte en commission : les principales dispositions ont été supprimées, sur la base d'arguments dont j'aurai l'occasion de discuter du bien-fondé.

Au mois de décembre dernier, après avoir annoncé un premier ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des Français, dispositions approuvées par la Haute Assemblée, le Président de la République a réuni à l'Élysée les représentants des mutuelles, des assureurs et des instituts de prévoyance. Comme aux grandes entreprises et aux banques, il leur a demandé de prendre part à la mobilisation pour l'urgence économique et sociale. Les dépenses de complémentaires santé font en effet partie des dépenses dites « contraintes », celles auxquelles les ménages ne peuvent échapper. Les organismes complémentaires ont répondu à cet appel et se sont engagés à prendre des mesures pour le pouvoir d'achat des assurés : la hausse des tarifs prévue en 2019 pour les contrats d'entrée de gamme devra être neutralisée, et les organismes complémentaires s'engageront dans un travail commun pour faire évoluer à la baisse les frais de gestion, qui représentent environ 20 % des cotisations collectées. En outre, l'une des propositions qu'a évoquées le Président de la République et que traduit cette proposition de loi est de faciliter les conditions de résiliation, donc de laisser plus de liberté aux ménages et de réduire les tarifs des complémentaires en faisant davantage jouer la concurrence. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai entendu les critiques qui ont été émises en commission et qui ne manqueront pas de s'exprimer au cours de ce débat, lors de l'examen des amendements de rétablissement. Ainsi, comme j'ai pu le faire à l'Assemblée nationale, je saisis l'occasion qui m'est offerte de m'exprimer à la tribune pour éclairer le débat et répondre à certaines idées reçues qui circulent sur ce texte.

D'ailleurs, la mise en oeuvre de mesures similaires dans d'autres secteurs de l'assurance ne s'est pas traduite par des hausses de primes, au contraire. Par exemple, la mise en oeuvre de la résiliation annuelle des contrats d'assurance emprunteur depuis le 1 janvier le 1 janvier 2018 a conduit certains organismes à diminuer leurs primes de 30 %. Ensuite, cette mesure ne va pas favoriser les comportements opportunistes.

Un assuré qui souhaiterait souscrire une complémentaire santé avant un acte médical programmé, puis s'en défaire après cet acte, ne pourrait donc pas mettre surcroît, cette mesure ne va pas déstabiliser le marché. Elle favorisera la mobilité des assurés qui souhaitent changer de complémentaire santé. Néanmoins, d'un point de vue global, elle ne modifiera pas drastiquement la situation actuelle, car une résiliation annuelle est déjà possible. Dès lors, chacun peut changer de contrat chaque année. J'ajoute que, au titre de la loi Hamon de 2014, l'on n'a pas identifié d'effet déstabilisateur. Enfin, cette mesure ne va pas entraîner une démutualisation des risques au détriment des personnes âgées. Les garanties en termes de mutualisation seront inchangées, y compris en faveur des plus vulnérables les mutuelles et les autres organismes proposant des contrats responsables, qui constituent la quasi-totalité des contrats, ne peuvent recueillir d'informations médicales auprès de leurs membres, ni fixer de cotisations en fonction de l'état de santé des assurés. Le risque de démutualisation avait déjà été brandi lors de la discussion de la loi Hamon, notamment pour ce qui concerne l'assurance emprunteur. Or il ne s'est pas concrétisé : les tarifs ont fortement diminué à l'avantage de tous, y compris des personnes en risque aggravé de santé.

Ce travail conjoint a donné lieu à des avancées majeures ; je pense à la réforme du 100 % santé, qui a été construite en lien étroit avec l'ensemble des acteurs, et en particulier avec les fédérations d'organismes complémentaires. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, même si son objet peut paraître circonscrit, cette proposition de loi est d'une grande importance c'est une mesure concrète, qui, en levant les obstacles actuels au changement de complémentaire santé, aura un réel impact sur le quotidien des Français.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'assurance maladie complémentaire couvre plus de 95 % de la population française et finance 13 % de notre dépense de santé, représentant ainsi 36 milliards d'euros de cotisations collectées. Essentielle pour l'accès aux soins, cette protection constitue un poste de dépense lourd pour les ménages, comme pour les entreprises qui participent au financement de la couverture collective, désormais généralisée, de leurs salariés. Les organismes privés qui opèrent pour l'essentiel sur ce secteur ont fait face ces dernières années à d'importantes mutations. Ils sont encore appelés à s'adapter, notamment pour contribuer aux efforts en faveur du pouvoir d'achat des Français,

Sans engager de révolution, elle suscite des réactions marquées, ce qui a conduit notre commission à en rejeter le dispositif central, en adoptant des amendements de nos collègues Philippe Mouiller et Jean-Marie Morisset. Le but initial de ce texte est clairement circonscrit : permettre aux assurés de résilier à tout moment leur contrat de complémentaire santé, après la première année de souscription. C'est, non pas une nouveauté, mais une souplesse donnée aux ménages comme aux entreprises.

mesure s'inscrit dans une tendance générale : la loi Hamon de 2014 a ouvert un droit à résiliation infra-annuelle pour les assurances auto et habitation. Dans un autre domaine, celui de l'assurance emprunteur, notre collègue Martial Bourquin a été à l'initiative d'une mesure visant à faciliter les résiliations de contrat.

inutilement les organismes, dans un environnement qui a déjà connu d'importantes restructurations. Du fait de la particularité de l'assurance en santé, ils craignent que le nomadisme n'entraîne des comportements opportunistes ou consuméristes susceptibles de porter atteinte aux mécanismes de mutualisation et de solidarité, au détriment des assurés les plus fragiles, notamment les plus âgés. La santé n'est pas un bien comme un autre. Nous en sommes tous intimement convaincus. Pour autant,

En toute honnêteté, il serait excessif de lui imputer une diminution significative des tarifs, que certains espèrent, ou une explosion des frais de gestion, que d'autres redoutent. elle porte sur un domaine tout à fait différent, la loi Hamon n'a pas eu de tel effet sur le secteur des assurances dommages, et nul ne songe aujourd'hui à revenir sur cette avancée. Si la santé n'est pas un bien comme les autres, le secteur de l'assurance complémentaire est bel et bien un marché. Ce simple constat n'emporte aucun jugement de valeur Sénat, nous sommes nombreux à régulièrement pointer du doigt l'insuffisante efficience de ses opérateurs, en appelant à une modération de leurs frais de gestion ou à une plus grande transparence. À mon sens, ce texte pourrait apporter une pierre à l'édifice : il contribuerait à créer les conditions d'un marché plus fluide, et les opérateurs auraient intérêt à proposer de meilleures garanties, au meilleur tarif. débat, la commission des affaires sociales a considéré que les dispositions introduites par ce texte soulevaient plus d'interrogations qu'elles n'apportaient de réponses. Elle a donc supprimé les articles 1, 2, 3 et 4 ouvrant la voie à la résiliation infra-annuelle des contrats santé proposés par les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles. Vous comprendrez que je regrette, à titre personnel, cette position. Néanmoins, au cours du débat, nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets, qui appellent- j'en conviens -des clarifications.

S'il est essentiel de sécuriser la mise en oeuvre du tiers payant en cas d'un plus grand turnover des contrats, le déploiement de services numériques par les organismes complémentaires doit s'accompagner de l'équipement des professionnels et établissements de santé en outils adaptés.

De même, en supprimant la demande de rapport destinée à évaluer les progrès accomplis quant à la lisibilité des contrats, la commission n'a pas entendu remettre en cause l'impérieuse nécessité de traduire en actions concrètes les engagements pris en ce début d'année par les organismes complémentaires. La complexité des garanties offertes, en partie inhérente à notre système, qui superpose deux niveaux de prise en charge, est un réel frein pour comparer les contrats et tarifs et permettre à la concurrence de s'exercer sainement.

de loi initiale vise à permettre aux assurés, particuliers comme entreprises, de résilier sans frais et à tout moment, après la première année de souscription, leur contrat de complémentaire santé, que celui-ci ait été signé avec une mutuelle, une assurance ou une institution de prévoyance. Après des velléités de présentation, sans concertation préalable, d'un amendement au titre du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, ou projet de loi Pacte,

cette proposition de loi apporte une mauvaise solution à un problème qui n'existe pas. Oh ! Aujourd'hui, personne n'est prisonnier de sa complémentaire santé. peut en changer chaque année, sans frais ; et chacun doit en changer, toujours sans frais, lorsqu'il change d'employeur, quand il est couvert dans le cadre d'un contrat de groupe. Un an de réserve, d'une part ; un an de visibilité, un an de garanties pour l'assuré, d'autre part : tel est le modèle prudentiel français de gestion. Dans ces conditions, s'agit-il d'améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens,

ne rémunèrent pas d'actionnaires, sont gérées à l'équilibre conformément aux exigences prudentielles liées aux risques, mettent en oeuvre des services qui accompagnent les adhérents tout au long de la vie et répartissent les risques entre les générations. L'évolution des cotisations est liée à celle des prestations. Le taux de la taxe de solidarité additionnelle, ou TSA, a été porté de 2,5 % à 13,27 % entre 2008 et 2012, et il est majoré de 0,8 % en 2019 en substitution au forfait patientèle.

La publicité et le marketing représentent 0,2 % du budget du mouvement mutualiste. Or l'adoption de la résiliation infra-annuelle ne pourrait qu'engendrer une hausse de ces frais de publicité, destinée à fidéliser les adhérents et à en conquérir de nouveaux.

Il est tout de même paradoxal de regretter un régime où la concurrence règne, avec, pour conséquence, des frais de publicité jugés excessifs et, dans le même temps, de vouloir mettre en place les conditions d'une concurrence totalement dérégulée.

en réduisant la complémentaire santé à un bien de consommation courante, pour lequel la seule question qui vaille est le calcul des coûts et des avantages pour soi-même, et rien que pour soi-même, le présent texte heurte le pilier de notre système de protection sociale : la valeur de solidarité. loi profitera peut-être à des assurés solvables, plutôt jeunes, actifs, bien portants, à faible risque, dans une logique purement assurantielle. Mais, en encourageant l'individualisation des risques accentuant la segmentation des populations, elle déstabilisera le principe de mutualisation, sur lequel le modèle économique des mutuelles est assis. Elle fragilisera encore un peu plus les mécanismes de la solidarité intergénérationnelle.

Couverts à 75 % par des mutuelles, ils bénéficient aujourd'hui de tarifs maîtrisés grâce aux mécanismes de solidarité que permet la mutualisation. En revanche, les jeunes seront encore plus fortement encouragés à individualiser leurs risques en se tournant vers les propositions les moins chères.

dans leur essence même, au modèle prudentiel français. Elles encouragent l'individualisation du droit au détriment de logiques collectives et universelles. Le risque de comportements opportunistes, consuméristes ou nomades sera bien sûr limité, mais non quand une partie importante des frais de santé pris en charge par les complémentaires correspondent à des dépenses programmables. Troisièmement, et enfin, cette proposition de loi, si elle est adoptée, sera un frein au développement du tiers payant. Grâce aux efforts de l'association Inter-AMC, créée en 2015 et regroupant tous les acteurs de la sphère complémentaire, quelque 83 % des assurés sont aujourd'hui couverts par des solutions techniques permettant aux professionnels de santé d'interroger en temps réel les droits et garanties garanties des assurés. Ainsi, les organismes complémentaires sont prêts à donner aux professionnels de santé des garanties de paiement, sur présentation d'une carte de tiers payant. Avec la résiliation possible à tout moment, le risque d'indus deviendrait évidemment difficile à maîtriser. C'est donc à raison que la commission des affaires sociales, le 10 avril dernier, a supprimé l'ensemble du texte issu de l'Assemblée nationale, à l'exception d'un article, l'article 3 , qui porte sur les informations données à l'assuré. En cohérence

nous avons déposé un amendement de suppression de l'article 3 AA, introduit en commission, qui interdit de moduler les remboursements selon que l'assuré s'adresse ou non à un professionnel appartenant au réseau de santé de son de son organisme de complémentaire santé. Je le rappelle rapidement : les réseaux de soins sont fondés sur des partenariats entre des mutuelles et des professionnels de santé qui s'engagent à respecter des critères de qualité

mes chers collègues, depuis 2010, les tarifs des complémentaires de santé augmentent de manière substantielle, et les frais de gestion représentent une part très importante des cotisations payées par les assurés. Forts de ce constat, les auteurs de cette proposition de loi ont souhaité assouplir le droit de résiliation et permettre aux assurés de bénéficier d'une concurrence accrue.

l'essentiel, cette proposition de loi se résume actuellement à deux mesures : la communication aux assurés du taux de redistribution des contrats et une disposition introduite en commission des affaires sociales, sur l'initiative de notre collègue Daniel Chasseing, visant à proscrire les pratiques de remboursement différencié. Notre groupe salue l'adoption de cette mesure. L'accès de tous les Français à des soins de qualité doit en effet être une priorité absolue. Permettre aux mutuelles d'opérer une différenciation dans le remboursement des prestations bouleverse les principes fondamentaux de notre modèle de santé, fondé sur la solidarité, la liberté et l'égalité dans la qualité de prise en charge. Le remboursement différencié remet en cause le principe « à cotisations égales, prestations égales », porte atteinte à la liberté de choix et de prescription et, enfin, accentue les inégalités territoriales. Pour en revenir au dispositif central du texte, dont nous aurons à débattre à l'occasion de l'examen des amendements, j'entends j'entends les griefs avancés, notamment, par les fédérations des complémentaires santé, lesquelles dénoncent « une fausse bonne idée qui aura un impact négatif pour les assurés » et sera « porteuse de risques majeurs ». Nous avons été

Comme l'a rappelé notre rapporteur en commission, il serait exagéré de penser que tous les particuliers et toutes les entreprises vont se saisir de cette nouvelle faculté. Il suffit d'observer les effets de la loi Hamon

L'objectif de ce texte est simple : faciliter la vie des assurés en leur apportant davantage de liberté et rééquilibrer le rapport de force en leur faveur. C'est la raison pour laquelle, avec plusieurs sénateurs du groupe du Rassemblement Démocratique au projet de loi Pacte visant à introduire un peu plus de concurrence, dans un contexte d'inflation des tarifs des complémentaires santé. Les chiffres communiqués par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la Drees, sont en effet édifiants : entre 2008 et 2017, les frais de gestion des complémentaires santé ont augmenté en moyenne de 4,2 % par an, soit deux fois plus vite que les dépenses de santé, pour atteindre 7,3 milliards d'euros. Cela représente 21 % du coût des cotisations, alors que le budget santé devient insupportable pour la plupart des ménages. La cotisation moyenne à une complémentaire santé s'élevait ainsi en 2017 à 688 euros par an, soit une progression trois fois plus rapide que l'inflation dans la dernière décennie. Cette situation n'est pas acceptable ! Aujourd'hui encore, bon nombre de Français sont contraints de se priver de soins en raison d'un reste à charge trop élevé, parce que leur couverture santé est souvent insuffisante. Les élus de la République ne peuvent y être indifférents. Je me félicite, enfin, que ce texte offre également l'occasion de simplifier les informations transmises aux assurés concernant le montant des frais de gestion, des prestations versées et des cotisations afférentes. Cette mesure, demandée à plusieurs reprises par des associations de défense des consommateurs, poursuit un objectif de transparence qui sera, j'en suis convaincu, bénéfique à l'ensemble des assurés.

Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à ouvrir le droit à résilier, sans frais ni pénalité, un contrat de complémentaire santé à tout moment, au-delà de la première année de souscription, et non plus seulement à la date d'échéance annuelle du contrat. Rien de plus ! Avant d'aborder le

donc un renforcement adapté de la prise en charge solidaire assurée par le premier niveau. Cependant, les salariés qui bénéficient obligatoirement d'une complémentaire négociée par leur employeur

risques. En créant deux types de contrats, les contrats collectifs et les contrats individuels, nous avons opéré par le passé une segmentation du marché, qui n'a pas pu se faire en faveur des retraités, tandis que les salariés voyaient leur couverture augmenter, sans que cela garantisse pour autant son adéquation à leurs besoins. En conclusion, dans la mesure où le législateur a souhaité imposer un panier de soins minimum aux contrats collectifs de santé, nous pouvons considérer que l'État a ouvertement voulu augmenter le niveau de prise en charge d'une grande partie de la population. Cela revient à faire peser sur le secteur privé un objectif de santé publique qui, étant déconnecté des besoins des individus, ne devrait relever que de la solidarité nationale, donc de la sécurité sociale. Dès lors, il aurait mieux, d'une part, valu revaloriser le niveau des remboursements de la sécurité sociale dans les domaines faisant partie du panier de soins minimal, et, d'autre part, rendre obligatoire pour tous les Français la souscription d'un contrat de complémentaire santé, tout en obligeant les OCAM à proposer un contrat d'entrée de gamme à très faible coût pour satisfaire ceux qui ne souhaitaient pas initialement en bénéficier. Madame la ministre, vous en êtes déjà convaincue, rien n'est plus intime que la santé ; nous avons tous nos spécificités et nos risques. Dès lors, puisque nous ne pouvons pas rendre la santé totalement gratuite, définissons clairement le niveau minimum de prise en charge qui devrait relever uniquement de la solidarité nationale et laissons à chacun la liberté d'adapter précisément sa couverture en fonction de ses besoins et de ses propres risques.

À titre personnel, et avec plusieurs de mes collègues, je soutiendrai la réintroduction des articles supprimés en commission, d'abord parce que l'extension des dispositions de la loi Hamon, entrée en vigueur le 1 janvier 2015, aux contrats complémentaires santé n'a rien de choquant juridiquement.

Enfin, la Cour des comptes elle-même déplorait que les OCAM aient dépensé 7,2 milliards d'euros en frais de gestion, dont près de 3 milliards d'euros en simples frais de publicité et de communication afin d'obtenir de nouveaux clients.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'amélioration du pouvoir d'achat est une des premières préoccupations des Français. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui visait, dans sa version initiale, à permettre la résiliation sans frais et à tout moment d'un contrat de complémentaire santé, après un an de souscription, de prévenir le nomadisme. Madame la ministre, il est prévu que tout changement de mutuelle soit bien notifié dans le dossier pharmaceutique du patient, afin de ne pas affecter le remboursement des pharmaciens qui pratiquent le tiers payant et dont les marges ont fortement diminué. Actuellement, les conditions de changement de mutuelle sont très strictes : un assuré ne peut résilier son contrat qu'en cas de changement de régime de sécurité sociale ou chaque année, à la date anniversaire de la souscription. Comme le souligne Michel Amiel dans son rapport, cette proposition de loi s'inscrivait dans une démarche globale de facilitation des conditions de résiliation des contrats d'assurance. Il s'agissait d'aligner le régime de résiliation des contrats de complémentaire santé sur les évolutions récentes issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, offrant la possibilité de résilier, après un an, les contrats d'assurance multirisque habitation, responsabilité civile et automobile. Ces évolutions visent à rendre du pouvoir d'achat aux Français en favorisant la concurrence et la liberté des assurés de résilier et de souscrire le contrat de leur choix, correspondant au correspondant au mieux à leur budget et à leurs besoins. Nous connaissons tous le rôle crucial des mutuelles dans le système de soins français. 95 % des Français ont recours à ce deuxième régime assurantiel, qui représente à lui seul 26 milliards d'euros, soit 14 % des dépenses de santé globales. Dans un contexte de vieillissement de la population et de forte augmentation de la prévalence des maladies chroniques, conjugué aux dépassements d'honoraires, en particulier dans les métropoles, l'accès aux complémentaires santé devient un élément incontournable pour garantir

financières à se soigner. Les trois millions de Français qui ne disposent pas d'une assurance maladie complémentaire sont les plus vulnérables. Nous le savons, dans une économie ouverte, les rigidités contractuelles sont susceptibles de freiner l'accès aux mutuelles des personnes les plus vulnérables économiquement. Notre groupe est donc favorable au rétablissement du texte. À l'heure où les dépenses de sécurité sociale sont amenées à être rationalisées, entraînant un report vers la prise en charge par les par les complémentaires, il apparaît légitime de demander aux mutuelles davantage d'efforts en faveur du pouvoir d'achat, car celles-ci disposent encore de marges de manoeuvre importantes pour normaliser leur fonctionnement. Les frais de gestion restent trop élevés, 20 % des cotisations, les règles de remboursement sont complexes pour l'assuré et les coûts des cotisations ont augmenté de 47 % dans la dernière décennie. Notre groupe avait déposé un amendement en commission visant à proscrire les pratiques de remboursement différencié au sein des réseaux de soin mis en place par les mutuelles. Nous saluons l'adoption de cette mesure, qui contribuera à garantir à chacun la liberté de choisir son professionnel de santé, en particulier dans les territoires ruraux sous-dotés en médecins. Madame la ministre, mes chers collègues, au cours de l'examen de ce texte, la majorité de notre groupe votera en faveur de la liberté contractuelle, dans la mesure où cela n'impacte pas le remboursement des professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant. Nous en appelons également à la sagesse de la Haute Assemblée et du Gouvernement pour maintenir la disposition adoptée par notre commission visant à proscrire les pratiques de remboursements différenciés par les complémentaires

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, s'il nous fallait aujourd'hui construire un système d'assurance maladie, il ne fait pas de doute que nous procéderions autrement nous ne ferions pas le choix de plusieurs traitements successifs d'un même acte, ce qui se traduit par des coûts de transaction élevés ; nous ne ferions pas le choix d'un système inégalitaire, dans lequel les mieux portants sont mieux couverts pour un coût moins élevé nous ne ferions pas le choix de la coexistence de quelque 500 organismes complémentaires en situation de concurrence. Notre système actuel à deux étages est le fruit de l'histoire, et, comme le Gouvernement en fait l'expérience en matière de retraite, la refonte globale d'un système présente bien des écueils, qu'aucun gouvernement n'a souhaité affronter en matière de santé. Les gouvernements successifs se sont pourtant essayés à la réforme, mais avec des objectifs peu clairs, des orientations pas toujours cohérentes et, sans surprise, des résultats mitigés.

Les contrats responsables encadrent le contenu des garanties, avec l'objectif d'agir sur les prix, en laissant peu de marges sur le contenu. La La fiscalité, levier fortement mobilisé, ponctionne une partie des profits réalisés, mais se retrouve dans les cotisations. le reste à charge zéro, on tente une reconquête de pans entiers de la couverture sociale, délaissés par le régime de base : l'optique, le dentaire, l'auditif, en encadrant davantage encore les complémentaires. Il résulte de ces différentes mesures un marché très administré, un corset réglementaire et fiscal sophistiqué, mais qui reste peu protecteur de ceux qui n'entrent dans aucun dispositif spécifique : les jeunes, les inactifs, les retraités. Très complexe, le système comprend de larges poches d'inefficience, alors que les besoins en matière de santé vont croissant et nécessitent de valoriser chaque euro disponible pour les défis qui sont devant nous : le vieillissement de la population, la chronicisation des maladies ou encore les innovations coûteuses. Avec cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, le Gouvernement privilégie un autre levier, celui du renforcement de la concurrence entre les acteurs, en assouplissant les possibilités de résiliation des contrats au-delà de l'actuelle possibilité de résiliation annuelle à la date anniversaire du contrat. L'évaluation de l'impact de cette mesure est difficile : baisse des coûts et hausse du pouvoir d'achat pour les uns, risque de nomadisme et de démutualisation pour les autres ; les débats ont été nourris, y compris ont été nourris, y compris au sein de la commission des affaires sociales. Il me semble peu probable que cette disposition bouleverse l'économie des contrats collectifs des grandes entreprises. Celles-ci ont les moyens de sélectionner au mieux l'organisme qui leur convient et de gérer leur calendrier de résiliation, par ailleurs enserré dans un processus de négociation collective. Pour les plus petites entreprises, comme pour les adhésions individuelles, le texte apporte une souplesse supplémentaire par rapport à la possibilité de résiliation annuelle. Comment les acteurs vont-ils s'en saisir et quelles vont en être les conséquences sur le marché ? Si l'on en croit les précédents, en particulier celui de la loi Hamon, le marché ne devrait pas s'en trouver bouleversé à l'excès, sans doute, que par les ratios de solvabilité imposés par les normes internationales ou par la mise en oeuvre du reste à charge zéro. Les cotisations ne devraient pas non plus baisser drastiquement sous l'effet de cette seule possibilité de résilier à tout moment. Au total, le texte soumis à notre examen me paraît renforcer les possibilités de choix de leur complémentaire santé pour les souscripteurs individuels, en particulier les retraités, et les petites entreprises. Il leur appartiendra de s'en saisir.

aux objectifs de ses fondateurs. Très bien ! Il faut donc opérer un décroisement des flux financiers au sein d'un ensemble devenu inextricable.

je voterai pour la possibilité, après douze mois d'affiliation, de résilier un contrat de complémentaire santé à tout moment. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dire que cette proposition de loi a eu un parcours tumultueux est un doux euphémisme. À l'origine, la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé devait être annoncée par le Président de la République dans le cadre des mesures d'urgence de décembre dernier, en réponse à la mobilisation des « gilets jaunes ». Puis, elle devait être intégrée au projet de loi Pacte. De crainte d'une censure du Conseil constitutionnel, elle a été reculée une seconde fois. C'est finalement le groupe La République En Marche, majoritaire à l'Assemblée nationale, qui a déposé ce projet de loi déguisé et l'a fait adopter, malgré les désaccords de plusieurs plusieurs députés de son propre camp. Au Sénat, la droite sénatoriale s'est livrée à une volte-face en quelques semaines. En effet, lors de la première réunion de la commission des affaires sociales, le groupe Les Républicains avait vertement critiqué cette possibilité de résiliation des contrats et avait voté la suppression des articles correspondants.

L'obstination du gouvernement auquel vous appartenez, madame la ministre, à la priver du principe des cotisations est, à ce titre, un véritable coup de boutoir ! Il s'agit aussi d'un recul pour toutes les personnes qui renoncent aux soins à cause du coût des contrats. Selon le comparateur des assurances, le coût annuel d'une mutuelle santé atteint 1 732 euros par an, en moyenne, pour un retraité, 981 euros pour les personnes à la recherche d'un emploi et 482 euros pour les étudiants. J'ajoute que la dernière publication de la Drees a chiffré à 4 millions le nombre de personnes non couvertes par une complémentaire santé, alors même que celles qui en sont dépourvues renoncent deux fois plus aux soins plus aux soins que les autres. Vous voulez nous faire croire qu'accroître la concurrence sur le marché de l'assurance complémentaire santé, en permettant de résilier sans frais et à tout moment les contrats, va diminuer leurs tarifs, mais c'est faux. Le marché- c'est dans sa nature ! -suit l'unique objectif de la rentabilité financière ; les effets bénéfiques en matière de baisse de tarifs sont donc rarement au rendez-vous, ou alors au prix d'une dégradation de la qualité des biens et des services. Nous avions d'ailleurs entendu le même discours lors de l'introduction d'un quatrième opérateur téléphonique. Finalement, les prix ont certes baissé, mais 10 000 emplois ont été détruits, et nous avons pris un retard considérable dans le déploiement du haut débit. La concurrence accrue entre les opérateurs à tout moment de l'année pourrait même s'avérer contre-productive, puisque les frais de gestion vont mécaniquement augmenter à cause d'un plus grand turnover dans les contrats des adhérents et de l'augmentation des frais de publicité. Cette offensive libérale va, de surcroît, affaiblir les principes mutualistes qui fondent notre protection sociale : la non-sélection du risque, l'égalité de traitement, la transparence, l'action sociale. En imposant des règles identiques aux instituts de prévoyance, aux assurances santé et aux mutuelles, vous allez encore accélérer le processus de rapprochement du mode de gestion des mutuelles à but non lucratif de celui des sociétés d'assurances à but lucratif. En ouvrant la possibilité de résilier un contrat au bout d'une année, vous remettez en cause le principe d'annualité des cotisations, un élément du modèle économique qui permet de ne sélectionner ni le risque couvert ni la personne. Demain, avec des contrats plus courts, il faudra segmenter davantage les populations en fonction de leurs risques spécifiques face à la maladie, et les seniors seront alors les grands perdants de la réforme. Dans un secteur de plus en plus concentré, votre texte ne fera que renforcer les mastodontes de la « bancassurance » pour faire primer le fonctionnement assurantiel sur la logique de solidarité.

complémentaires risque, selon nous, d'accroître les inégalités sociales dans l'accès aux soins. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette proposition de loi.

Un cap, puisqu'elle vise à redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens ; un souffle, puisqu'elle entraîne les mutuelles dans un cercle économique plus vertueux ; une stratégie, parce que, dans sa conception première, elle répond à nombre de problématiques et elle accompagne le mouvement engagé par le reste à charge zéro. Je me réjouis de voir que, à l'issue d'un travail de commission remarquablement argumenté par notre rapporteur, vous avez enfin identifié le cap qu'elle prenait, le souffle qu'elle suscitait et la stratégie qu'elle développait. Avant tout, je tiens à remercier mon collègue et ami, Michel Amiel, rapporteur de ce texte, de la qualité du travail réalisé dans des délais très restreints. L'objectif de ce texte, il l'a rappelé, est simple : donner la possibilité aux assurés de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription leurs contrats de complémentaire santé. N'oublions pas ce qui sous-tend ce texte : l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages par la réduction des dépenses contraintes pesant sur les familles et, plus encore, sur les plus fragiles et les plus précaires. Cette proposition de loi s'inscrit dans une action globale menée par le gouvernement et dans le mouvement engagé par la réforme du reste à charge zéro sur les soins dentaires, optiques et auditifs. Aujourd'hui, nous nous emparons d'un nouveau volet : le coût de la complémentaire santé, qui doit être adapté aux besoins de nos concitoyens.

Sur la base d'un millier d'échéanciers pour 2019, l'UFC-Que Choisir a également dénoncé une progression des tarifs entre 2018 et 2019 de près de 8 % en moyenne, l'augmentation pouvant aller jusqu'à 25 % pour certains contrats. Avec l'adoption de cette proposition de loi, l'économie pour les consommateurs pourrait atteindre 1 milliard d'euros par an. Simplifier les démarches et améliorer le pouvoir d'achat sans remettre en cause la solidarité entre les assurés : tel est l'objectif du texte. texte. Aussi suis-je heureux de constater aujourd'hui que les esprits ont évolué, preuve que la sagesse du Sénat n'est pas un vain mot

! ... la rédaction proposée par le rapporteur, qui rejoint celle du Gouvernement, reste pour moi la meilleure, car elle protège davantage l'assuré.

37 % des Français trouvent leur garantie santé difficile à comprendre et 48 % d'entre eux ne connaissent pas à l'avance, pour les soins importants, le montant du remboursement qu'ils percevront.

en rétablissant le formalisme de la lettre recommandée en cas de résiliation sur l'initiative de l'assureur ou dans d'autres cas sujets à contentieux. Vous avez fait preuve d'un certain panache en revenant sur vos décisions en commission.

texte affirment de manière péremptoire que cette mesure « donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé ». On croirait un mauvais slogan des années on lit également que, « compte tenu de l'ampleur des montants versés chaque année au titre des cotisations en matière d'assurance santé- 35,9 milliards d'euros en 2016 -, la proposition de loi vise à accroître la concurrence sur le marché de l'assurance complémentaire santé Pourtant, il n'y a aucun lien logique, d'après moi, entre le volume annuel des cotisations et l'accroissement souhaité de la concurrence. De la même manière, on avance des chiffres au sujet de l'augmentation des tarifs des complémentaires santé entre 2018 et 2019,

de résiliations, ayant pourtant entraîné des frais de gestion relativement importants pour les compagnies d'assurances et,, les particuliers. Résultat, les cotisations de l'assurance dommages des particuliers n'ont pas diminué

quelque 80 % des cotisations sont reversées en prestations et 20 % paient les frais de gestion, alors que ceux de la sécurité sociale sont inférieurs à 4 %.

Depuis plusieurs années, l'État fait le choix de diminuer le niveau des prestations de santé ou la prise en charge. En conséquence, les remboursements en frais médicaux de la sécurité sociale ont diminué, tandis que les frais pris en charge par les complémentaires santé ont augmenté.

Que faut-il en déduire ? D'un côté, on cherche l'intérêt du consommateur en lui permettant de résilier à tout moment sa complémentaire santé et de mener une guerre des prix pour gagner du pouvoir d'achat ; de l'autre, dans le même texte, on souhaite la suppression des réseaux de santé, qui ont pourtant prouvé qu'ils limitaient les coûts de santé et amélioraient le pouvoir d'achat des bénéficiaires

n'est même pas un marché du tout ... Il serait dangereux de déstabiliser le principe de solidarité qui prévaut dans notre société. Si tel est le chemin que nous voulons emprunter, pour une raison ou pour une autre, réfléchissons de manière globale !

n° 15 rectifié. L'article 2 de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les institutions

d'abord, à rétablir le formalisme de la lettre recommandée- chose importante -en cas de résiliation sur l'initiative de l'assureur ou dans d'autres cas sujets à contentieux ; ensuite, à opérer des harmonisations rédactionnelles avec la terminologie retenue par l'ordonnance de 2017 sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier ; enfin, à supprimer certaines formulations ambiguës. La parole

eux. La lettre recommandée et l'envoi recommandé électronique apportent la sécurité juridique de l'acte, s'agissant surtout des dates précises de souscription des contrats. L'assureur devra maintenant confirmer par écrit la réception de la notification de résiliation : cela créera de nouveaux contentieux et des frais supplémentaires, qui seront encore comparés aux frais de gestion de la sécurité sociale. C'est pourquoi le présent sous-amendement tend à supprimer les dispositions introduites à l'Assemblée nationale relatives aux modalités de résiliation. Le sous-amendement n° 8, présenté

en rétablissant le formalisme de l'envoi recommandé dans plusieurs situations sources de contentieux. D'autres assouplissements pouvaient paraître justifiés dans une perspective de simplification.

la question de l'extension du droit à résiliation infra-annuelle aux contrats de prévoyance se pose en effet, mais les enjeux financiers sont lourds, notamment pour les entreprises qui proposent ces garanties à leurs salariés, de façon souvent concomitante avec les contrats de complémentaire santé.

Accroître la concurrence dans le domaine de l'assurance complémentaire santé revient à s'en remettre au marché pour assurer l'égal accès aux soins. Or, contrairement à ce que prétendent les chantres du libéralisme économique, la santé n'est pas une marchandise Accroître la concurrence entre les acteurs de la santé n'est donc absolument pas gage d'une amélioration de l'accès aux soins, bien au contraire. Ce texte va renforcer les mastodontes de la « bancassurance », pour faire prévaloir le fonctionnement assurantiel sur la logique de solidarité et développer des contrats de santé low cost. vous mettez fin au principe de la redistribution entre bien portants et malades et entre riches et pauvres, au profit d'une logique d'individualisation des risques en fonction de l'âge, de l'état de santé et des habitudes de vie de chacun. En réalité, le Gouvernement refuse de s'attaquer au vrai problème : les inégalités d'accès aux soins dans notre pays. Si vous aviez réellement voulu réduire le reste à charge des assurés, madame la ministre, il fallait diminuer les taxes sur les contrats de complémentaire santé, au lieu de les augmenter.

cette concurrence risque au contraire de laisser de côté les plus fragiles et de mettre à mal notre système de solidarité intergénérationnelle. Elle risque de se traduire par une guerre entre complémentaires pour capter les assurés, au détriment de la qualité des contrats proposés. Ce texte a été l'occasion pour certains de montrer du doigt le fonctionnement des OCAM, au vu notamment de leurs frais de gestion démesurés, disproportionnés par rapport à ceux de l'assurance maladie obligatoire. Il faut mesurer que l'assurance maladie obligatoire, comme il n'a pas à sa charge la perception des cotisations. Par ailleurs, elle n'est pas taxée à hauteur de 13,27 % et n'est pas soumise à la réglementation européenne, non plus qu'à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur les salaires. Madame le ministre, vous le savez bien l'évolution des primes d'assurance et des frais de gestion est due principalement au poids des réformes réglementaires annuelles et à l'augmentation des dépenses de santé et du prix des médicaments.

et se sont inscrits dans une synergie avec les autorités publiques. Pourquoi donc leur imposer une double peine, en les obligeant à modifier de nouveau leurs règles de gestion pour s'adapter aux conséquences concrètes de cette

Deuxième observation, cette proposition, quoi que l'on puisse en dire, remet bien en cause l'un des fondements du financement des actes médicaux et des frais de santé, à savoir la présomption de couverture en cas de présentation d'une carte d'adhérent à une complémentaire santé. Cette mesure, je l'ai déjà dit, mais c'est important, ne facilitera pas le développement du tiers payant. Troisième observation, l'un de nos collègues a souligné le caractère symbolique de ce texte. Oui, il s'agit d'un symbole très fort. C'est le triomphe de la concurrence comme philosophie de la protection sociale ! Or nous sommes nombreux à penser que la solidarité n'est pas soluble dans la concurrence ou dans les logiques de court terme- beaucoup se sont exprimés sur ce point.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

du Sénat sur l'action du Gouvernement. Madame la ministre, les chaînes d'information sont aujourd'hui mobilisées en boucle sur l'affaire de la Pitié-Salpêtrière.

Très vite, des témoignages contraires ont montré que nous étions peut-être en face d'un mouvement de panique, des personnes voulant simplement s'enfuir et se protéger

n° 15 rectifié. L'article 2 de la proposition de loi, supprimé par la commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. Cet amendement vise à rétablir cet article, qui constituait, avec les articles 1 et 3, également supprimés, le coeur du dispositif de la proposition de loi. Il apporte des ajustements à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en procédant à des harmonisations rédactionnelles ou à la suppression de mentions ambiguës et en rétablissant le formalisme de la lettre recommandée dans certains cas qui sont sujets à contentieux.

nous ne sommes pas les seuls ! Les institutions de prévoyance et la mutualité française ont fait part des risques d'augmentation des coûts de gestion et, par conséquent, des tarifs des contrats. Les cinq confédérations syndicales vous ont adressé la ministre, pour dénoncer un dispositif qui va à l'encontre de la liberté de négociation collective d'entreprise et de branche. Les associations de patients vous

contre-productif et dangereux pour l'accès aux soins des plus précaires. Madame la ministre, lorsque tant de personnes de sensibilités politiques diverses et aux responsabilités différentes

de cette création majeure. Si le temps qui s'est écoulé a vu la mise en concurrence faire son oeuvre, l'Union européenne rapprochant le fonctionnement des mutuelles de celui des assurances en niant les principes démocratiques et non lucratifs du mutualisme, il n'en demeure pas moins que les principes mutualistes

vous allez fragiliser la mutualisation sur laquelle repose le modèle économique des mutuelles. D'autre part, vous allez accroître le nomadisme médical : la seule question qui se posera alors sera celle du rapport coût-avantage pour soi-même, et rien que pour soi-même. Or, si les jeunes pourront individualiser leurs risques en se tournant vers les complémentaires santé les moins chères et offrant les couvertures les moins étendues, généralement proposées par les « bancassurances », nos aînés, eux,

la profession concernée. Comme l'indique l'Autorité de la concurrence, les réseaux ont un effet bénéfique sur les marchés concernés, tant pour les professionnels de santé affiliés que pour les assurés, même s'agissant des réseaux fermés.

une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé. En effet, les réseaux de soins qui existaient déjà n'étaient ouverts qu'aux organismes de prévoyance et aux sociétés d'assurance, et non aux mutuelles. Il fallait donc les ouvrir à l'ensemble des organismes complémentaires, mais aussi les encadrer, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, des inspections générales des finances et des affaires sociales, et ce afin d'améliorer l'accès aux soins. Nous avons donc encadré le dispositif, qui ne l'était pas du tout, en garantissant le libre choix du professionnel ou de l'établissement par le patient, des critères objectifs, transparents et non discriminatoires pour l'adhésion du professionnel ou de l'établissement à la convention, et l'interdiction de toute clause d'exclusivité. Nous avons également proposé- c'est très important -d'exclure du conventionnement tous les actes médicaux bénéficiant d'un tarif conventionnel de la sécurité sociale, quel que soit le professionnel. Aujourd'hui, les réseaux de soins font, à nos yeux, l'objet d'une attaque injustifiée en matière d'accès aux soins, alors que la question de fond réside dans la désertification médicale. Ne leur faisons pas porter une responsabilité qu'ils n'ont pas

des équipements. Or, selon l'IGAS, le recours au réseau permet de réduire de 46 % le reste à charge moyen sur l'achat de deux verres pour adultes, par exemple. C'est pourquoi le groupe socialiste fera preuve

des potentiels adhérents et souscripteurs, qui est imposée aux organismes assureurs, a pour objectif d'aider les consommateurs à effectuer un choix éclairé. C'est pourquoi cette information doit être, d'une part, intelligible et compréhensible, et, d'autre part, uniformément présentée par les différents organismes assureurs, de façon à faciliter la comparaison.

a pour objet de préciser que ces deux ratios doivent être présentés hors taxes, comme c'est le cas actuellement, de sorte que les éventuelles modifications de la fiscalité sur les contrats d'assurance ne viennent pas perturber l'information des assurés. L'amendement n° 6 rectifié,

dès le 1janvier 2020.

La République En Marche. Il a été décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Alain Richard, auteur des propositions de loi. Monsieur

une série d'observations, pour porter à la connaissance du public et, naturellement, des autres pouvoirs publics les améliorations qu'il conviendrait d'apporter au droit électoral, ou, d'ailleurs, à d'autres sujets connexes de droit public. C'est

et dont les montants de dépenses paraissaient négligeables. Nous avons essayé, dans la proposition de loi, d'établir un tel critère, afin de pouvoir identifier les candidats « minimaux », dirais-je, auxquels serait accordée une dispense de compte de campagne, ce qui réduirait la charge de travail des institutions en aval. Le Conseil constitutionnel faisait également remarquer, à l'observation de ses propres décisions individuelles, que, du fait de la durée des contentieux, une même même sanction d'inéligibilité- deux ans par exemple -portant sur des infractions ou des manquements de même importance n'avait pas les mêmes conséquences pour deux candidats différents, suivant que la date d'expiration de la période d'inéligibilité englobait l'élection suivante ou non.

on limite le terme final des réunions électorales au vendredi soir, comme pour les autres actes de campagne. Enfin, constatant que la jurisprudence, aussi bien du Conseil d'État, pour les élections locales, que du Conseil constitutionnel, pour les élections parlementaires,

ce qui est tout de même un peu décalé par rapport à l'objet même du bulletin de vote, lequel est, non plus un outil de communication, mais un support du vote le plus objectif possible -, il nous a paru souhaitable d'éliminer, par la loi, la référence à des personnes tierces, non candidates dans la circonscription,

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, notre éminent collègue Alain Richard, qui vient de s'exprimer, de s'exprimer, nous invite à clarifier diverses dispositions du code électoral, qui, depuis 1956, a effectivement perdu en lisibilité et en cohérence, malgré les tentatives d'harmonisation de la Commission supérieure de codification. Nul doute que la présence la présence de dispositions de valeur organique a constitué un obstacle. La proposition de loi et la proposition de loi organique s'inspirent assez directement des observations rendues par le Conseil constitutionnel le 21 février dernier au sujet des élections législatives

d'une part, clarifier le contrôle des comptes de campagne et les règles d'inéligibilité ; d'autre part, mieux encadrer la propagande électorale et les opérations de vote. Au cours de ses travaux, la commission des lois a salué ces efforts de clarification. Ces textes auront des conséquences concrètes, notamment pour simplifier les démarches administratives des candidats et mettre fin à certains détournements de procédure en matière de propagande électorale. Les nombreux amendements déposés ont démontré tout l'intérêt de ces véhicules législatifs, à la fois techniques et transversaux. Notre collègue Alain Richard propose, tout d'abord, de simplifier les démarches administratives des candidats et d'améliorer les contrôles de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques- Nous constatons effectivement une massification du contentieux, qui complique les contrôles, de l'aveu même du Conseil constitutionnel et de la CNCCFP. Lors des élections législatives de 2017, le nombre de candidats ayant déposé un compte de campagne a augmenté de 27 % par rapport au scrutin précédent. En conséquence, la commission nationale a saisi le juge de l'élection à 351 reprises, soit une hausse de près de 50 % par rapport à 2012. Pour les élections départementales de 2015, elle a contrôlé plus de 9 000 comptes de campagne, avec des moyens qui sont reconnus comme limités. Je rappelle qu'elle dispose de 39 agents permanents et recourt à quelques rapporteurs vacataires, qu'elle s'adjoint au gré des élections. élections. Contrairement à la préconisation initiale du Conseil constitutionnel, la commission des lois n'a pas souhaité modifier le périmètre des comptes de campagne, craignant de fragiliser les contrôles de la CNCCFP. Elle Elle a privilégié d'autres mesures pour alléger les démarches administratives des candidats, notamment en élargissant la dispense d'expertise comptable. Aujourd'hui, seuls les candidats dont le compte ne comprend aucune recette ni dépense sont dispensés de recourir à un expert-comptable. sachez que, lors des élections législatives de 2017, plus de 3,5 millions d'euros ont servi à rémunérer des experts-comptables, ce qui représente près de 5 % des dépenses électorales Le texte de la commission élargit la dispense d'expertise-comptable aux candidats qui remplissent deux conditions cumulatives : d'une part, s'ils ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ; d'autre part, si leurs recettes et leurs dépenses n'excèdent pas un montant fixé par décret. Entendu en audition, l'ordre des experts-comptables ne s'oppose pas- bien au contraire -à cette simplification, considérant que le chiffre d'affaires de ses membres ne dépend pas de cette intervention, qu'il qualifie de « devoir citoyen Des amendements de nos collègues Roger Karoutchi et Josiane Costes nous inciteront à aller plus loin dans nos démarches de simplification, notamment en ce qui concerne les « menues dépenses » des candidats. Notre collègue Jean-Pierre Grand nous propose, avec l'appui du Gouvernement, d'autoriser les candidats à recourir aux plateformes en ligne pour recueillir des dons. Demande forte des candidats, cette mesure nécessitait de nombreuses garanties, notamment pour assurer la traçabilité des dons ; le Gouvernement nous les apporte. En complément, la commission des lois a adopté plusieurs mesures techniques, notamment pour mieux organiser les contrôles de la CNCCFP et confirmer l'interdiction, pour les personnes morales, d'apporter leur garantie aux prêts contractés par les candidats. la proposition de loi organique visent également à clarifier les règles d'inéligibilité. Aujourd'hui, en effet, le code électoral distingue plusieurs hypothèses d'inéligibilité, ce qui affecte sa lisibilité. En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales par le candidat ou si celui-ci n'a pas déposé son compte de campagne, le juge « peut » prononcer l'inéligibilité. En revanche, il a l'obligation de déclarer inéligible un candidat « dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales En pratique, et nous aurons certainement ce débat ultérieurement, à l'occasion de l'examen d'un des amendements, le juge prononce l'inéligibilité seulement lorsqu'il estime que l'irrégularité constatée présente un degré de gravité suffisant.

Pour plus de lisibilité, les présents textes tendent donc à clarifier le rôle du juge en mettant en accord le code électoral et la jurisprudence, comme l'a d'ailleurs préconisé le Conseil constitutionnel. Je le rappelle avec force à cette tribune, il ne s'agit en aucun cas d'affaiblir le régime des inéligibilités, qui doit s'appliquer avec la plus grande fermeté à l'encontre des candidats fautifs. Il y va de la crédibilité de notre système institutionnel. En commission, nous avons eu un débat concernant le « point de départ » de l'inéligibilité. Aujourd'hui, cette sanction s'applique à compter de la décision définitive du juge de l'élection. Tout le monde s'accorde sur les inconvénients de cette disposition : pour une irrégularité équivalente, à l'autre, en fonction du délai d'instruction de l'affaire. Initialement, la proposition de loi et la proposition de loi organique tendaient à faire démarrer l'inéligibilité à la date du premier tour de scrutin. Cette solution présentait toutefois plusieurs inconvénients.

Dans une volonté de compromis, la commission des lois a proposé un dispositif alternatif, qui lui a semblé plus équitable. Le juge électoral sera invité à moduler la durée des inéligibilités prononcées, afin que les candidats ayant commis des irrégularités comparables

La commission a également clarifié l'inéligibilité prononcée contre les parlementaires pour manquement à leurs obligations fiscales, notamment pour confirmer que les fautifs ont l'interdiction, pendant la durée de leur inéligibilité, de se présenter à d'autres scrutins.

S'agissant des bulletins de vote, il est proposé d'y interdire l'apposition de la photographie ou de la représentation des tierces personnes, mais également du candidat ou de son suppléant. Étonnamment, le Conseil constitutionnel avait admis, dans une décision rendue en décembre 2017, la représentation sur un bulletin de vote aux élections législatives d'une tierce personne, maire d'une commune et ancien député de la circonscription, alors que cela pouvait

que nous avons tous apprécié à différentes occasions, permettra d'éviter les accusations de « tambouille électorale ». Le pouvoir réglementaire sera tenu de respecter cette règle,

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 21 février, le Conseil constitutionnel a rendu une décision dans laquelle il fait part de ses observations relatives aux dernières élections législatives. Cette décision était riche d'enseignements et de propositions pour améliorer notre droit électoral. effectivement, et vous le savez bien en qualité d'élus, que le droit électoral recèle parfois de petites zones d'ombre involontaires, qui peuvent semer le trouble chez les électeurs, mais aussi chez les candidats, et poser des difficultés au juge électoral.

Ainsi, en l'état du droit, et du fait d'une divergence entre la partie législative et la partie réglementaire du code électoral, la tenue de réunions publiques est possible la veille du scrutin, tandis que la distribution de matériel électoral, le collage d'affiches ou l'émission de messages électoraux dans les médias ou sur les réseaux sociaux sont interdits depuis le vendredi soir, à minuit, ou le samedi matin, à zéro heure.

les actes. L'autre grande avancée permise par ce texte consiste à rendre toute leur sincérité aux bulletins de vote. La loi interdit déjà de faire figurer sur un bulletin de vote le nom d'une personne qui ne s'est pas portée candidate. Cependant, cette interdiction fait l'objet d'une jurisprudence assez permissive. Grâce à ce texte, nous avons l'occasion de remettre les choses en place. Ainsi, l'interdiction de faire mention du nom d'un tiers sur un bulletin de vote est explicitement renforcée au travers de cette proposition de loi. Cela évitera des détournements ou des pièges pour les électeurs.

un terme à de telles démarches, en interdisant formellement la présence de photos ou de représentations autres que celles des candidats sur leurs bulletins de vote. à souligner que la proposition de loi d'Alain Richard permet bien d'autres progrès pour notre loi électorale, y compris en dehors des recommandations émises par le Conseil constitutionnel. Je pense, en particulier, aux précisions sur les délais et la qualité de la déclaration de situation de patrimoine à produire pour prétendre au remboursement des frais de campagne. Le code électoral était jusqu'ici trop flou et cette proposition de loi règle la question, en se fondant sur les propositions de la Haute Autorité

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'adaptation des règles électorales aux difficultés ou évolutions constatées lors de leur mise en oeuvre est toujours utile pour la vitalité démocratique. Lorsque les fonctions électives sont fragilisées, comme on le constate aujourd'hui, cette adaptation devient impérative. En ce sens, l'initiative de notre collègue Alain Richard, prise à la suite de la publication, en février dernier, des observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017, est particulièrement bienvenue. Il faut d'ailleurs souligner sa grande réactivité. Les membres du groupe du RDSE regrettent que le pouvoir réglementaire ne mette pas autant d'ardeur à prendre des décrets d'application une fois la loi adoptée L'ensemble des modifications proposées, qu'il s'agisse de la simplification des règles comptables s'appliquant aux candidats, de la clarification des règles de propagande électorale ou encore de l'adaptation du point de départ des des décisions d'inéligibilité aux réalités des procédures contentieuses, nous semblent aller dans le bon sens. Les amendements introduits par notre rapporteur modifient certains points techniques des deux propositions de loi, sans en trahir l'esprit. C'est pourquoi nous sommes favorables à leur adoption. En effet, chacun conviendra ici que l'annulation d'une élection par le juge n'est jamais satisfaisante, laissant planer une ombre de discrédit sur l'ensemble des élus. Pour autant, cette initiative rappelle à nos concitoyens que les candidats à une élection s'exposent à une grande insécurité juridique, du fait de la complexité des règles électorales, mais aussi de l'incertitude liée à l'issue du scrutin, conditionnant les obligations qui leur seront applicables. C'est, par exemple, le cas des règles de contrôle des comptes de campagne. Dès lors qu'une dérogation existe au-dessous du seuil de 1 %, selon les règles actuelles, on comprend que des petits candidats, ayant peu d'espoir sur l'issue du scrutin, ne prennent pas toutes les précautions nécessaires pour se mettre en règle, tant ces régularisations comportent un coût non négligeable. D'autres notions, aux contours mal définis, car strictement jurisprudentiels, comme celle de « dépense électorale », rendent plus incertaine leur aptitude à se conformer aux règles en vigueur. Notre collègue Josiane Costes a d'ailleurs déposé des amendements de clarification en ce sens. Ainsi, les irrégularités constatées par le juge sont moins révélatrices de la faible moralité des candidats que de la complexité des règles applicables. Certains vont même jusqu'à considérer que ces règles forment une barrière d'entrée décourageante pour les candidats les moins bien conseillés, et qu'elles accaparent une partie du temps qu'ils pourraient mettre utilement à profit pour l'élaboration de propositions au contact de leurs électeurs. Elles sont cependant incontournables dans le cadre d'un financement en majorité public de la vie politique française, dès lors que tout engagement de deniers publics doit être justifié. Leur renforcement, depuis 1995, a d'ailleurs pour objectif d'assainir le financement de notre vie démocratique et de prévenir l'influence de puissances financières ou étrangères sur l'issue des suffrages. De nombreux États européens disposent d'ailleurs d'une législation comparable et ont été amenés à en renforcer la transparence, sous l'influence notable du Conseil de l'Europe. plusieurs voix s'élèvent contre le régime de financement actuel, pour proposer des systèmes alternatifs comme, par exemple, la création d'une « banque de la démocratie » ou le passage à un financement strictement privé et transparent comme au Royaume-Uni., au Royaume-Uni., d'autres proposent le renforcement du financement public, avec un rapprochement de l'encadrement des dons des particuliers, considérant que, dans leur écrasante majorité, les Français n'ont pas les moyens de donner 7 500 euros à la formation politique de leur choix. Une réflexion globale sur le sujet, monsieur le ministre, pourrait s'engager en parallèle de la réforme des institutions en cours de préparation. Ce questionnement est légitime, car, comme l'estiment certains économistes, le financement de la vie politique coûterait 32 euros par an à chaque Français, par le biais des impôts. la nécessité de simplification et d'adaptation du code électoral à l'évolution des attentes de nos concitoyens dépasse les seules dispositions du texte adopté par la commission des lois, le grand nombre d'amendements déposés pour la séance. C'est peut-être le seul regret que nous exprimons à ce stade : la grande réactivité de notre collègue ne nous permet pas de conduire un travail de toilettage Cette initiative aurait par exemple pu être l'occasion d'analyser les défauts de l'encadrement du cumul des mandats, en particulier le sort des suppléants : aucune disposition n'a été prévue pour que ceux-ci retrouvent leurs fonctions initiales à la fin de leur suppléance. Les amendements de notre collègue Jean-Pierre Corbisez visent également à alerter sur les « candidats TGV », c'est-à-dire ceux qui participent à des élections sur des territoires avec lesquels ils n'ont aucun lien effectif ou affectif. Le phénomène est actuellement rendu possible par la trop grande panoplie des pièces admises pour prouver sa résidence dans une commune par les services de l'État. me permet de rappeler les défaillances du contrôle préfectoral sur l'organisation des élections, problème sur lequel le groupe du RDSE a déjà insisté par le passé. contrôle ne sera pas renforcé, il sera plus difficile de faire respecter les décisions d'inéligibilité ou la suspension du droit de vote pour les personnes dont l'altération de l'entendement a été reconnue par une décision d'incapacité. Enfin, lors de l'examen de ce texte, certains amendements pourraient nous faire revenir sur notre position favorable s'ils étaient adoptés. Je pense par exemple à celui qui a pour objet de modifier la règle de découpage des circonscriptions électorales, amendement rejeté en commission.

les règles de financement de la vie politique, notamment des campagnes électorales. Je salue la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Elle découle d'observations du Conseil constitutionnel. Elle vise à clarifier en apportant de la cohérence aux dispositions du droit électoral, notamment celles qui concernent les comptes de campagne et la propagande électorale. L'agrégat de dispositions pour le moins sédimentées au sein du code électoral, modifiées au fil du temps sans véritable réflexion globale, a affaibli la lisibilité et la cohérence des procédures électorales. En effet, depuis 2011, sept lois ont modifié le chapitre relatif au financement et au plafonnement des dépenses électorales. Les démarches administratives complexes créées par cet enchevêtrement juridique posent d'autant plus problème que le nombre de candidats ayant dû déposer un compte de campagne est en hausse notable. De ce fait- cela a été rappelé -, le risque de contentieux s'est accru, et les instances chargées du contrôle sont en surrégime. Je salue ainsi la proposition du rapporteur dispensant les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages et dont les recettes et dépenses n'excèdent pas un certain montant de recourir à un expert-comptable. Une telle obligation peut en effet se révéler inutile et excessivement coûteuse, sans être

Il reviendra au juge de prononcer l'inéligibilité lorsque les comptes seront rejetés « à bon droit », en cas de manquement d'une particulière gravité ou de volonté de frauder. Il ne s'agit donc plus d'une obligation. Cette marge d'appréciation permettra ainsi au juge de ne pas prononcer l'inéligibilité pour des erreurs vénielles.

le délai d'instruction varie d'un dossier à l'autre, avec l'engorgement lié à la hausse des contentieux. Ainsi, un candidat dont le dossier aura été instruit très rapidement pourra avoir la possibilité de se présenter au scrutin suivant, ce qui n'est pas le cas de celui dont le jugement ne sera prononcé que quelques mois plus tard. Je salue donc la proposition du rapporteur visant à moduler la durée de l'inéligibilité, notamment au regard du calendrier électoral, afin de garantir une équité entre deux ou plusieurs candidats en situation similaire. Une autre incohérence existe à ce jour. Il est possible de faire une réunion publique la veille de l'élection jusqu'à minuit, mais pas de distribuer le moindre document de propagande

ni nom d'une tierce personne, nous semble aller dans le bon sens, afin d'éviter d'induire les électeurs en erreur, parfois d'une manière lourde, mais peu visible. Vous l'avez compris, le groupe Union Centriste estime que les dispositions de cette proposition de loi sont positives,

le ministre, mes chers collègues, le code électoral, qui fut créé en 1956, a été conçu comme un instrument de clarification à destination des électeurs et des candidats. Réunissant les modes de scrutin des élections locales et parlementaires, il s'est substitué à plus de quatre-vingt-dix textes éparpillés et sans cohérence. Sa structure n'a pas été revue depuis, malgré les tentatives de la Commission supérieure de codification, à la fin des années 2000. En outre, la présence de dispositions de valeur organique exclut tout recours aux ordonnances, outil privilégié pour créer de nouveaux codes ou les réorganiser. Le code électoral rassemble ainsi des articles récents, en voie de sédimentation, et des dispositions très anciennes, comme celle qui renvoie encore aux lois fondatrices de la III République. Sans revoir l'ensemble de ce code, les deux textes de notre collègue Alain Richard ont deux objectifs : d'une part, ils clarifient le contrôle des comptes de campagne et les règles d'inéligibilité ; d'autre part, ils encadrent mieux la propagande électorale, ainsi que les opérations de vote. Ils s'inspirent directement des observations formulées par le Conseil constitutionnel sur les élections législatives de 2017. Toutefois, ils concernent l'ensemble des élections, y compris les élections locales. Je me réjouis tout particulièrement des efforts de clarification de ces textes, qui ont été enrichis par la suite en commission des lois par diverses mesures d'ordre technique. viens au contrôle des dépenses électorales. La commission n'a pas souhaité modifier le périmètre des comptes de campagne, craignant de fragiliser les contrôles de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Je me félicite qu'elle ait privilégié d'autres mesures pour alléger les démarches administratives des candidats, comme l'élargissement de la dispense de recourir à un expert-comptable. La commission des lois a également veillé à assurer une certaine équité entre les candidats déclarés inéligibles sans modifier le point de départ de l'inéligibilité. Ainsi, le juge électoral serait invité à moduler la durée des inéligibilités prononcées, afin que les candidats ayant commis des irrégularités comparables soient déclarés inéligibles pour les mêmes échéances électorales ; cela a été très bien souligné par le rapporteur. En matière matière de propagande, la commission a admis l'interdiction d'organiser des réunions électorales la veille de l'élection, et plus seulement le jour du scrutin, notamment pour répondre au risque de contentieux et sécuriser la campagne des candidats.

De même, elle a interdit les publicités à caractère commercial dans les six mois qui précèdent le scrutin. Elle a mieux encadré le contenu des bulletins de vote, notamment pour interdire l'apposition d'une photographie et la mention d'une tierce personne. Enfin, la commission des lois a inscrit dans le code électoral la tradition républicaine selon laquelle les règles électorales ne sont pas modifiées dans l'année qui précède le scrutin.

les deux propositions de loi en discussion visent à rénover plusieurs aspects du droit électoral. Cette initiative correspond à un besoin bien identifié de clarification, d'actualisation et de lisibilité de la norme électorale. La commission des lois du Sénat l'avait déjà souligné en 2011, dans un rapport d'information relatif à l'évolution de la législation applicable aux campagnes électorales déposé, entre autres, par nos collègues Jean-Pierre Vial et Yves Détraigne. Il est vrai que, par leur technicité et leur champ restreint, les détails de la loi électorale ne sont pas de prime abord les sujets qui font l'objet de grands débats parmi nos concitoyens. Néanmoins, cette norme est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Une loi électorale claire, équitable et efficace renforce la confiance des citoyens envers leurs élus et le processus démocratique dans son ensemble. C'est aussi dans cet esprit que la codification des normes électorales a été effectuée en 1956. Ces normes ont beaucoup évolué depuis lors, ce qui rend tout à fait légitime un effort de mise à jour. C'est donc avec une attention toute particulière que nous examinons les deux propositions de loi, qui oeuvrent en ce sens. La diversité des enjeux pratiques, juridiques et démocratiques abordés n'en fait pas pour autant un inventaire à la Prévert. Ces textes portent sur des questions importantes : dépenses électorales, règles d'inéligibilité et propagande électorale. D'une part, la proposition de loi organique concerne tout particulièrement l'inéligibilité des parlementaires nationaux et les questions financières. Elle simplifie certaines rédactions et renforce l'importance de la notion de « volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales Des amendements de la commission ont également remanié un dispositif destiné à permettre au juge de moduler la durée des inéligibilités en fonction du calendrier électoral, afin de faire en sorte que les durées variables des procédures ne conduisent pas à des inégalités entre candidats justiciables ; tout cela a été fort bien expliqué. D'autre part, la proposition de loi ordinaire s'inscrit dans la même logique de consolidation et de simplification du droit électoral. Tout comme la proposition de loi organique, elle contient des mesures relatives au financement des campagnes électorales. Sans revenir sur l'ensemble des dispositions, parfois relativement techniques, je mentionne l'élargissement de la dispense d'expertise-comptable aux candidats ayant obtenu moins de 5 % des voix et l'harmonisation du délai d'instruction devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. D'autres dispositions concernant la propagande électorale et les opérations de vote viennent également corriger certaines incohérences et lacunes. Ainsi, il résulte d'une loi de 1881 que des réunions électorales peuvent encore se tenir la veille du scrutin à l'exclusion de toute autre manifestation ou distribution de matériel de propagande. L'article 4 de la proposition de loi aligne ce régime sur celui des autres formes de propagande, tandis que l'article 5 explicite les dispositions du code électoral relatives au contenu à inscrire, et à ne pas inscrire, sur les bulletins de vote. Dans cette même logique, l'article 5 , ajouté par la commission, clarifie certaines règles de propagande plus spécifiques aux élections sénatoriales, pour lesquelles un certain risque de contentieux a pu être identifié. Enfin, le texte propose également de consacrer au plan législatif le principe de stabilité du droit électoral durant l'année précédant le scrutin. Ce principe, qui relevait jusqu'ici de la tradition républicaine, s'appliquerait à l'ensemble des élections, à l'exception de l'élection présidentielle. Toutes ces mesures reflètent un travail fouillé et sérieux de clarification et de simplification. Ces textes devraient contribuer à une plus grande clarté du droit électoral tout en le consolidant là où se trouvaient des lacunes. En oeuvrant ainsi à l'amélioration de la qualité de la norme électorale, le Sénat inscrit également son action en cohérence avec les préconisations et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en effet évoqué en 2017 la modulation de la durée des inéligibilités, afin de limiter les inégalités entre candidats.

Premier exemple de simplification : la dispense de l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages. Je défendrai un amendement tendant à étendre cette disposition aux candidats qui, ayant obtenu moins de 5

En réglant le problème, nous pourrons limiter les dégâts. Un autre exemple de simplification et clarification est beaucoup plus intéressant et important pour moi : la suppression de l'automaticité de la peine d'inéligibilité qui existe actuellement pour certains types de manquements seulement. N'en déplaise aux moralistes impénitents, cette disposition me semble d'autant plus judicieuse que l'évaluation des comptes de campagne est loin d'être une science exacte, comme on va le voir. D'abord, le volume des dossiers à examiner dans le temps d'examen imposé ne met pas la CNCCFP à l'abri des erreurs et des approximations Ainsi, lors des élections législatives de 2017, elle a dû contrôler 5 427 comptes de campagne en l'espace de six mois, l'examen des cas ayant fait l'objet d'une saisine du juge électoral étant traité en deux mois.

un labyrinthe dans lequel se perdent beaucoup de candidats, malgré les trente pages du guide du candidat et du mandataire. Ainsi, le déjeuner d'une équipe de campagne ne constitue pas une dépense électorale, car il n'a pas d'effet direct sur les électeurs. À l'inverse, si l'équipe de campagne invite un journaliste à sa table, la dépense doit être déclarée à la CNCCFP. Côté recettes, les « concours en nature » sont particulièrement difficiles à cerner. Les services rendus à titre gratuit par des militants ne sont pas intégrés au compte de campagne, mais il faut prendre en considération leurs frais de déplacement, ainsi que leur action lorsqu'elle est en « lien direct » avec leur activité professionnelle. Autre problème : lorsqu'une entreprise casse ses prix, s'agit-il d'un simple rabais, alors légal, au profit d'un candidat ou d'un don d'une personne morale, La CNCCFP admet des rabais commerciaux allant jusqu'à 20 % du prix du marché. Mais comment calculer ce dernier, notamment dans le secteur de la communication ? du projet de loi de finances pour 2019, le président de la CNCCFP m'a confirmé que le coût des prestations de communication évoluait substantiellement en fonction du moment de la campagne, du délai de livraison et des éventuelles économies d'échelle même problème s'agissant de l'évaluation des marges facturées par les « ensembliers » qui organisent les meetings tout en faisant appel à des centaines de sous-traitants dont les factures ne sont communiquées ni aux candidats ni à la Commission. Lors de la dernière élection présidentielle, pour la première fois, la CNCCFP a eu recours à des experts- cela a été évoqué -pour évaluer les dépenses de campagne dans différents domaines : la seule chose sur laquelle ils se sont accordés, c'est qu'il était impossible de définir un prix du marché pour certaines prestations

Réponse du Conseil constitutionnel en 1995 : quelle que soit la grosseur des irrégularités, il vaut mieux valider le compte sans aller plus loin. C'est donc le compte de Jacques Cheminade qui a été rejeté, avec ce que cela signifie d'ennuis pour lui

pour un candidat à l'élection présidentielle de 2012 dont le compte de campagne avait été rejeté pour dépassement du plafond des dépenses électorales. Pourtant, elle le fait dans d'autres circonstances ... Au final, la proposition d'Alain Richard me paraît donc sage. À la CNCCFP de juger de la régularité de comptes de campagne difficiles à établir avec certitude : elle le fait honnêtement, avec les moyens dont elle dispose et les risques inhérents à ce genre d'exercice. Au juge le pouvoir de décider si des suites pénales doivent être données aux infractions constatées et, si oui, lesquelles. Ce n'est que prudence et justice. C'est pour cela que le groupe CRCE votera en faveur de cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 1898, le député Charles Ferry pouvait s'exclamer : « Pourquoi, après cinquante ans d'exercice constant du droit électoral sous la forme actuelle, inventez-vous [ ...] toutes ces chinoiseries ? » Le code électoral, ce sont toutes ces « chinoiseries » qui permettent d'organiser la compétition politique et, en démocratie, de garantir l'expression libre du suffrage, consacrée par l'article 3 de la Constitution. Cette expression libre se fonde, bien entendu, sur les principes d'égalité devant le suffrage, à la fois des candidats et des électeurs, et de sincérité du scrutin, lequel renvoie notamment aux conditions de financement des partis politiques et des campagnes électorales. Les deux textes que nous examinons aujourd'hui touchent donc à deux sujets d'autant plus fondamentaux qu'ils sont d'actualité : la démocratie et l'égalité. Ils s'appuient, comme cela a été dit, sur les observations du Conseil constitutionnel de 2017, qui reprennent d'ailleurs celles qui avaient été émises à l'occasion des élections législatives de 2012. double objectif : d'une part, clarifier le contrôle des dépenses électorales et les règles d'inéligibilité ; d'autre part, apporter des correctifs pour mieux encadrer la propagande électorale et les opérations de vote. Si nous souscrivons aux modifications proposées pour répondre à ce deuxième objectif, nous sommes beaucoup plus réservés sur celles qui sont relatives au prononcé de l'inéligibilité. Il y a bien, dans ces propositions, des correctifs utiles en matière de propagande électorale et d'opérations de vote.

La clarification apportée à l'article 5 au sujet du contenu du bulletin de vote revêt une importance certaine. Entre 1848 et 1913, la normalisation des bulletins de vote

un bulletin de vote. C'était aussi un moyen pour exprimer sa position sociale. Très vite, une standardisation a été instaurée, pas uniquement pour les bulletins de vote, mais pour l'ensemble des biens d'équipement politique : l'urne, l'isoloir, la feuille d'émargement, la disposition du bureau de vote, etc. Cette Cette codification montre tout simplement l'effort de rationalisation de l'État au cours de l'histoire et une volonté de mettre en place des instruments privilégiant l'égalité démocratique. La permanence de la possibilité de distinctions sur les bulletins nous semble donc problématique. Par ailleurs, elle ne participe pas à l'optimisation de la dépense publique, ce qui, historiquement, a été un motif pour l'État de standardisation, puisque le bulletin de vote est à sa charge. charge. Je veux signaler un autre point, probablement inattendu, à propos de la transposition dans le domaine législatif de la mention exclusive du nom du candidat, de son suppléant et du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant concerné.

proposé d'inscrire la mention : « en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité » en préambule du nouveau régime de cette sanction. Il appartiendra donc demain au juge de prouver cette volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité, alors qu'il n'a pas à le faire

la sanction. En vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. cause. Eu égard à cette jurisprudence, la proposition de loi constitue, selon nous, une remise en cause inutile des règles en matière de transparence et de financement de la vie politique.

En outre, s'il s'orientait vers des dispositions moins répressives et une proportionnalité de la sanction dans ses précédentes observations, le Conseil constitutionnel a aussi proposé d'autres modalités de sa saisine par la CNCCFP, en s'appuyant sur une inversion du contentieux.

Permettez-moi de m'étonner de cette proposition. En effet, si les candidats à une élection ne méritent aucun opprobre, ils ne doivent pas pour autant bénéficier de règles spécifiques. À ce titre, la proposition nous surprend de la part d'un de la part d'un parti politique qui a fait de l'exemplarité des élus sa marque de fabrique, sinon un argument de campagne. Et un article de presse récent titrait : « Loi électorale : les sénateurs s'arrangent avec les préconisations du Conseil constitutionnel ».

le symbole est fort, mais sans commune mesure avec les dispositions proposées. Pour conclure, si cette proposition de loi apporte, c'est vrai, des correctifs utiles, elle remet en question des règles de transparence et manque d'ambition sur la vie électorale et politique, alors même que le chef de l'État nous promet la mise en

On pourrait tout autant évoquer le financement de la démocratie, lequel reste profondément inégalitaire : la banque de la démocratie n'a finalement jamais vu le jour pour des motifs, il est vrai, soulignés par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi qui l'a instaurée, ce qui n'a pas empêché le Gouvernement de faire légiférer le Parlement en la matière. Les pouvoirs d'injonction du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques restent, quant à eux, mineurs puisqu'ils avaient notamment été pensés par rapport à cette banque de la démocratie qui n'a pas été mise en place. Pour toutes ces raisons, nous réservons notre vote à l'issue de l'examen de cette proposition de loi ; mais les articles relatifs à l'inéligibilité font, en tout état de cause, obstacle à un vote favorable de notre part. La parole

Roger Karoutchi. À la suite des élections législatives de juin 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi pour la première fois de la question suivante : un candidat peut-il valablement recevoir des dons par l'intermédiaire de l'opérateur de paiement en ligne PayPal Il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers, même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier. Il est proposé d'assouplir les dispositions en vigueur en permettant le recours à une telle modalité moderne de recueil de dons par les candidats et en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer un cadre garantissant

l'on en dispense les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, dont les recettes et les dépenses n'excèdent pas un montant fixé par décret.

que le candidat puisse régler directement de menues dépenses lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond

et ne facilite pas son application scrupuleuse. C'est pourquoi il est proposé de réfléchir à une définition plus précise et à l'établissement d'une liste qui pourrait être régulièrement actualisée par le Conseil d'État. Quel est l'avis de la commission ? Je salue cette ambition

la clarification de l'écriture ne change en rien le pouvoir du juge. Il n'y a absolument pas de recul, je le redis fortement.

En réalité, ce qui a malencontreusement été introduit dans le texte relatif aux pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière d'irrégularités faisant présumer une volonté frauduleuse prévoit une obligation de sanction.

en imaginant que le juge devrait automatiquement constater une volonté de fraude. Apprécier une volonté de fraude revient forcément à exercer un pouvoir juridictionnel. Le Conseil constitutionnel n'a par conséquent fait que nous rappeler que la législation antérieure était mal faite, qu'elle simulait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

? Sans vouloir encourager les agissements qui sont dénoncés et qui font l'objet des préoccupations de Roger Karoutchi, la commission a émis un avis défavorable sur cet

a pour objet de renforcer le lien effectif entre un candidat à une élection et le territoire sur lequel il se présente. Il est clair que nos règles en la matière doivent rester relativement flexibles, afin de permettre aux citoyens français attachés à différents territoires de vivre leur engagement politique dans celui de leur choix. C'est par exemple le cas de ce qu'on appelle les « conseillers forains qui choisissent de s'engager politiquement sur le territoire de leur résidence secondaire plutôt que sur le lieu de leur résidence principale. Il ne nous appartient pas de juger ce choix qui relève souvent plus de l'affect que d'autres considérations. Nous devons en revanche nous prémunir de certaines logiques opportunistes qui consisteraient à présenter des candidats sans aucun rapport avec la circonscription concernée. Ces stratégies contribuent à altérer les liens entre électeurs et élus, les électeurs pouvant à juste titre se sentir floués par de tels comportements. Elles dégradent également la qualité des campagnes électorales, en faisant passer le débat d'idées et de programme au second plan, après celui du débat d'éligibilité. Elles sont pourtant tolérées du fait de l'appréciation large par les services de l'État des pièces de nature à prouver l'inscription du candidat au rôle des contributions directes. Ainsi, un simple bail suffit, quand le candidat fait valoir que sa non-inscription au rôle est imputable à l'absence de diligence en ce sens de son bailleur. C'est pourquoi il est proposé de fixer le principe simple selon lequel on ne peut être candidat que dans le territoire où l'on est également électeur, afin de lutter contre le phénomène dit des candidats TGV, comme je vous l'avais déjà expliqué lors de la discussion générale. L'amendement

est l'un des principes de la loi de décentralisation de 1982. La commission a estimé normal que des citoyens qui entretiennent, et qui souhaitent continuer à le faire, des liens étroits avec une commune puissent s'y présenter, même s'ils n'y habitent pas. Les amendements

Lors des élections municipales, les préfets sont inéligibles dans le ressort où ils exercent pour une durée de trois ans ; ce délai de carence est d'un an pour les sous-préfets.

les affiches sont le dernier espace de liberté totale : c'est là où les candidats peuvent s'exprimer de manière libre. Pourquoi cette exception ? Tout simplement pour qu'on ne confonde pas les affiches des candidats avec les affiches officielles. pourquoi se priver de cette grande liberté que certains savent utiliser avec talent, dès lors que l'on sait que le juge intervient si les éléments figurant sur l'affiche induisent induisent les électeurs en erreur ? Nul doute que chacun a pu voter pour son député et n'envisageait pas d'envoyer siéger à l'Assemblée nationale le Président de la République, fut-il François Mitterrand, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron ... Quel est

voix l'amendement n° 37 rectifié. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que les présentes proposition de loi et proposition de loi organique ont été inscrites par la conférence des présidents dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe La République En Marche, c'est-à-dire pour une durée de quatre heures. Ce laps de temps étant écoulé, je me vois dans l'obligation d'interrompre l'examen de ces textes. Il reviendra à la conférence des présidents d'inscrire la suite de leur discussion à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.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

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, selon une estimation de la Banque mondiale, la corruption transnationale ferait perdre chaque année aux pays en développement entre 20 et 40 milliards de dollars, soit 20 % à 40 % du montant de l'aide annuelle au développement au plan mondial. La loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a élargi le champ des biens pouvant être saisis et confisqués, et créé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'Agrasc, qui assure la gestion des biens saisis et procède ensuite à leur aliénation. chers collègues, la convention des Nations unies contre la corruption prévoit la restitution obligatoire et intégrale des avoirs illicites au profit de l'État étranger victime dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits.

doit restituer les biens confisqués à l'État signataire requérant lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur ». Or ces règles sont rarement appliquées. En effet, elles n'entrent en vigueur que lorsque les juridictions étrangères ont engagé et mené à leur terme les procédures judiciaires nécessaires aux fins de recouvrer les avoirs illicites se trouvant à l'étranger. Par ailleurs, dans les cas de corruption transnationale et tout particulièrement lorsque les agissements illicites mettent en cause des agents publics de haut rang, parfois encore en exercice, il paraît souvent illusoire d'espérer que les États concernés rétrocèdent aux populations victimes le fruit de ces confiscations. Ainsi, la confiscation des produits de la corruption transnationale se trouvant en France emporte le plus souvent le transfert de leur propriété à l'État français. Quel est le but de la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter, mes chers collègues ? l'argent qui leur a été volé par la corruption internationale et par les agissements de toutes ces personnes, notables ou non, mais souvent déjà très riches,

et ce au mépris des populations qui ont été volées. Nous considérons que la situation en France est contraire à la pratique d'un nombre croissant d'États,

: garantir que les avoirs illicites recouvrés en France contribuent au développement des pays qui en ont été injustement privés et conforter les efforts de notre pays en matière de lutte contre la corruption transnationale dans tous les cas où l'absence de gouvernance ou l'état de défaillance des États d'origine rendent légalement impossible la mise en jeu des règles de partage ou de restitution. Transparency International ainsi qu'un certain nombre d'ONG, dont je tiens à saluer tout particulièrement l'action, proposent que, dans le dispositif d'affectation, cinq grands principes soient respectés la transparence- la procédure doit être conduite de manière publique ; la solidarité quant à l'affectation des fonds ; l'efficacité- il faut que l'argent revienne aux populations victimes

été privés. Il indique que « ces sommes blanchies, au lieu de financer des infrastructures et des services publics en Guinée équatoriale, étaient placées ou dépensées en France pour alimenter le train de vie particulièrement fastueux

l'État dont le président a aussi gravement fauté bénéficiait de ces sommes, il y aurait également un problème. C'est pourquoi le tribunal correctionnel de Paris affirme qu'il « paraît vraisemblable que le régime français des peines de confiscation

porte atteinte aux droits des populations concernées et représente le scandale et le comportement honteux des personnes qui s'enrichissent sur le dos d'êtres humains, qui sont souvent dans la situation la plus critique et la plus misérable.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur Jean-Pierre Sueur, auteur de la présente proposition de loi, mes chers collègues, aujourd'hui, lorsque la justice prononce la confiscation d'un bien, le produit de celle-ci revient au budget général de l'État, après une éventuelle indemnisation des parties civiles. Cette affectation à l'État français est moralement difficile à admettre lorsque les biens confisqués sont issus de la corruption dont profitent certains personnages de haut rang au détriment de leur population,

La proposition de loi de notre collègue que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans ce contexte ; il s'agit de proposer un cadre juridique permettant de rendre aux populations victimes de la corruption les confiscations prononcées par les juridictions françaises dans les affaires dites des biens mal acquis.

Ainsi, l'article 1 de la proposition de loi prévoit d'affecter les sommes concernées à « l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l'État de droit ainsi qu'à la lutte contre la corruption » dans le pays victime. On se heurte ici à la principale difficulté, d'ordre pratique : à qui doit-on effectivement affecter ces sommes ? À l'État, au risque d'alimenter de nouveau les circuits de corruption ? En outre, des États faillis ? Comment associer les acteurs locaux et contrôler l'utilisation des fonds ? Enfin, comment articuler de tels programmes avec notre action diplomatique ? Ces questions ne sont pas théoriques, comme le montre le cas récent de la saisie de biens appartenant à l'oncle de Bachar el-Assad : si des confiscations étaient prononcées par la justice française dans cette affaire, comment s'assurerait-on de l'affectation de leur produit à la population syrienne ?

Il pourrait être envisagé de s'appuyer sur l'Agence française de développement, compétente en matière d'aide au développement. Toutefois, il conviendrait de s'assurer que les crédits reviennent bien aux pays victimes sans être noyés dans ceux de l'Agence et, surtout, qu'il s'agit bien de crédits s'ajoutant à ceux qui sont engagés par la France au titre de l'aide publique au développement.

Ensuite, il conviendrait de déterminer le rôle joué par l'Agrasc dans cette procédure ; si l'Agence est capable d'identifier les confiscations devant être reversées aux populations victimes, elle n'est pas nécessairement l'institution la mieux à même de décider des modalités d'affectation à ces dernières, car elle n'a pas de compétences propres en matière d'aide au développement. Enfin, la commission des finances a émis des doutes sur la mécanique budgétaire retenue. Le prochain G7 sera organisé cet été à Biarritz, sous présidence française, et il traitera, entre autres, des moyens de lutter contre la corruption. Dans ce contexte, malgré les problèmes posés par le texte qui nous est soumis, il nous semble important d'envoyer un signal politique fort, indiquant que notre pays est prêt à s'engager à restituer aux populations victimes le produit des confiscations résultant de la corruption.

à la frontière du droit, de l'éthique et de la diplomatie : l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale- ces fameux biens dits « mal acquis » -et saisis par une juridiction française.

Pour lutter contre ce phénomène criminel à dimension transnationale, elle est également dotée, depuis 2010, d'une législation et de structures interministérielles dédiées à identifier, à saisir, à confisquer et à recouvrer des avoirs illicites, en particulier issus de la corruption. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'Agrasc, est précisément chargée de l'exécution des décisions de saisie et de confiscation, ainsi que de la gestion et de la vente des avoirs criminels confisqués. La France a par ailleurs créé tous les outils et mécanismes destinés à promouvoir, à développer et à appuyer la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption- c'est également un engagement fort de notre présidence du G7, vous l'avez rappelé ce qui constitue un volet clé pour récupérer, effectivement et rapidement, les fonds détournés ou soustraits illégalement du patrimoine d'un État. Cette politique nationale offensive s'inscrit donc pleinement

par des dirigeants ou des agents publics corrompus. L'état du droit ne permet pas la restitution de ces biens, sauf dans le cas d'un acte de souveraineté, qui prendrait la forme d'un accord politique entre la France et un pays tiers- accord difficile, reconnaissons-le, quand il s'agit des situations que vous avez décrites. Par conséquent, lorsqu'une décision de confiscation a été prononcée par une juridiction française, l'Agrasc n'a pas d'autre possibilité juridique que de transférer les fonds correspondants au budget général de l'État. Le droit français prévoit également une règle de partage à cinquante-cinquante, sauf accord contraire, lorsque la France est sollicitée pour exécuter une décision prise par une juridiction étrangère.

victimes de la corruption qui s'est d'abord faite à leur détriment, ne peuvent ensuite récupérer les sommes et les biens détournés par les dirigeants peu scrupuleux. Cette situation, je le répète, ne nous satisfait pas

De surcroît, les règles internationales en la matière évoluent. La convention des Nations unies contre la corruption, ratifiée par la France en 2005, prévoit la restitution obligatoire et intégrale des avoirs illicites au profit de l'État étranger. ses stipulations ne s'appliquent que très rarement, lorsque les juridictions nationales de l'État spolié ont mené à terme les procédures judiciaires nécessaires pour recouvrer les avoirs illicites dans la plupart des cas, les juridictions de l'État d'origine n'engagent pas ce type de demande, par crainte de représailles ou parce qu'elles ne le souhaitent pas pour toute autre raison. Plusieurs organisations de la société civile de premier rang, comme Transparency International, ont d'ailleurs souligné l'importance de la question du retour des biens mal acquis, en invitant les États à modifier leur législation.

J'ai ainsi appris que l'Allemagne avait mis en place, en 2017, un dispositif de restitution sans jugement préalable ; l'Italie permet de transférer des biens confisqués directement aux victimes

C'est dans ce contexte que nous examinons votre proposition de loi, cher Jean-Pierre Sueur. Je tiens à saluer de nouveau la très grande qualité de votre travail et les échanges que nous avons eus sur ce sujet délicat.

Le dépôt et l'examen de cette proposition de loi remplissent en ce sens pleinement leur office ; en interpellant l'ensemble des ministères concernés par cette difficile question, ce texte nous prépare d'ores et déjà à y apporter une solution. Notre ambition partagée doit être de restituer aux populations victimes les avoirs issus de la corruption, selon un mécanisme exigeant, précis, opérationnel et et permettant d'articuler différentes compétences, à commencer par celles de l'Agrasc, qui gère les avoirs saisis et confisqués et qui doit pouvoir identifier, sans ambiguïté juridique, l'ensemble des dossiers et des biens concernés. Cela suppose de définir un champ d'application rigoureux, concernant la nature tant des infractions que des personnes visées. Il faut également articuler ce mécanisme avec les services de l'État dépositaires d'une compétence et d'une expertise reconnues en matière d'aide au développement,

-qui permettent d'atteindre les objectifs politiques, humanitaires, sociaux et économiques que nous aurons. À cet égard, la présente proposition de loi crée un fonds destiné à recueillir les recettes provenant des confiscations prononcées en matière de corruption transnationale.

La première difficulté tient à la question cruciale de la répartition des compétences que j'évoquais à l'instant. Si un fonds devait être créé et alimenté par l'Agrasc, il resterait encore à en définir le positionnement et le cadre de gestion, compte tenu de sa finalité singulière. n'aurait en effet rien de comparable avec les fonds de concours déjà gérés par l'Agrasc, qui sont tous orientés vers le financement de politiques publiques nationales visant à renforcer la lutte contre la délinquance et la criminalité.

De la même manière, la notion de « personnes étrangères politiquement exposées » n'existe pas en droit pénal ; elle reste donc assez vague, et nous pouvons nous demander si elle permettra d'identifier réellement les personnes que nous souhaitons viser. Troisième difficulté- cela a été soulevé en commission -, les aspects relatifs au droit budgétaire et financier posent également problème, puisque la décision de créer un fonds au sein du budget général de l'État et de lui affecter des recettes relève du domaine exclusif de la loi de finances et non de celui d'une loi ordinaire. Enfin, il serait nécessaire d'expertiser davantage le montage juridique. Le financement d'actions de développement par le biais de l'affectation de recettes provenant de confiscations, comme le prévoit la proposition de loi, serait tributaire de l'avancée, par construction irrégulière,

qui feraient correspondre aux saisies en matière de corruption des dépenses équivalentes de développement. Que propose donc aujourd'hui le Gouvernement pour que le Parlement adopte un mécanisme de restitution efficace, transparent et adapté à chaque cas d'espèce ? D'abord, Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, lancera dans quelques jours une mission parlementaire sur le sujet précis, spécifique, du retour des biens mal acquis. Cette mission aura pour objet de proposer un mécanisme global traitant l'ensemble des difficultés juridiques, budgétaires et de gestion que j'ai rappelées et respectant les principes posés par la convention des Nations unies contre la corruption. Elle devra en particulier étudier chacune des pistes budgétaires qui sont aujourd'hui sur la table. Elle sera bien sûr utilement éclairée par les dispositifs mis en oeuvre par d'autres États.

Ce travail d'expertise complémentaire s'inscrira dans un calendrier très resserré, et le rapport de la mission sera remis au garde des sceaux au mois de juillet prochain. Il pourra s'appuyer utilement sur les travaux menés par la Haute Assemblée.

Nos engagements juridiques et diplomatiques, mais également nos valeurs et les principes républicains que nous défendons nous intiment d'y apporter enfin une réponse efficace. Vous l'aurez compris, cette réponse ne peut pas être celle que la commission des finances présente aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il ne pourra pas émettre un avis favorable sur cette version du texte.

Marc. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

La corruption transnationale renvoie à l'accaparement de biens publics ou privés au profit d'une minorité d'oligarques, qui bénéficient indûment d'un enrichissement illicite. Cette forme de corruption se caractérise notamment par les conséquences économiques et sociales injustes qu'elle fait peser sur les pays d'origine. Rappelons les chiffres de la Banque mondiale : chaque année, la corruption transnationale ferait perdre entre

Ce sont des pays qui se retrouvent ainsi privés des ressources dont ils manquent déjà pour financer leur développement de façon pérenne. Cette mécanique n'a, hélas, rien de nouveau, et l'argent qui est volé là-bas finit parfois par être investi ici. ici. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, mes chers collègues, nous fait envisager le problème sous un angle nouveau ; quand l'État fait respecter ici la loi et saisit ces biens mal acquis, il ne permet pas leur retour dans le pays d'origine, et il freine ainsi le développement économique et social Nul ne peut se satisfaire de cette situation, dans laquelle notre droit entérine de fait la spoliation de ces populations et échoue à indemniser les victimes de la corruption. C'est à cette fin que la France a ratifié, en 2005, la convention des Nations unies contre la corruption, qui fixe le cadre international de la restitution des avoirs confisqués à la suite de condamnations en matière de corruption. Des mesures ont déjà été prises dans notre pays pour appliquer cette convention, avec la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Mais cela ne suffit pas et nous devons encore poursuivre nos efforts dans ce sens, afin de donner corps aux engagements que nous avons pris sur la scène internationale. Au-delà de nos frontières, la Suisse a déjà fait bouger les lignes. Les premiers Les premiers retours d'expérience, recueillis après le traitement de plusieurs affaires symboliques, montrent que l'on peut agir pour tenter de réparer le dommage subi par les populations spoliées. manifestement d'un exemple intéressant. Cependant, derrière une intention noble se cachent de nombreuses difficultés pratiques. Premièrement, dans beaucoup de cas, il serait mal avisé de restituer ces biens confisqués à un État que nous savons défaillant. Deuxièmement, comment s'appuyer sur la société civile pour restituer à ces populations les ressources dont elles ont été spoliées ? Comment choisir un acteur privé pour lui confier une telle mission d'intérêt général ? Ici encore, l'exemple suisse nous montre qu'il n'existe pas de solution miracle et que chaque situation doit être traitée au cas par cas. Mais avant même de rencontrer ces difficultés que nous concevons lorsque nous envisageons le meilleur moyen d'agir par-delà nos frontières, nous nous heurtons à une première difficulté juridique. Comme l'a souligné le rapporteur, la création d'un fonds dédié au sein du budget de l'État, comme le prévoit la proposition de loi, ne paraît pas répondre aux prescriptions de la LOLF en matière d'affectation de recettes.

La solution appartient donc aujourd'hui au Gouvernement. Le groupe les Indépendants - République et Territoires suivra la position de la commission des finances et votera en faveur de l'esprit de la proposition de loi, en espérant que le Gouvernement se saisisse de l'appel que nous lui lançons aujourd'hui pour agir demain en matière de corruption transnationale.

Posons les termes : la corruption transnationale est le fait d'offrir un avantage indu, pécuniaire ou autre, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché dans le commerce international. Avec l'entrée en vigueur de la convention sur la lutte contre la corruption, la France a adopté plusieurs incriminations de corruption et de trafic d'influence en relation avec des agents publics étrangers. Elle a aussi étendu les pouvoirs des enquêteurs.

détournement de fonds publics et corruption commis en Guinée équatoriale. Elle a validé la vente des biens saisis et l'affectation de son produit au budget de l'État. Voilà où se situe la proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur Sueur : l'affectation des recettes provenant de la confiscation des sommes ou biens issus de la corruption aux populations des États où la corruption a eu lieu. Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués seraient ainsi affectés à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l'État de droit, ainsi qu'à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions en cause ont été Mon groupe s'abstiendra sur ce texte, car plusieurs points doivent encore être éclaircis. Tout d'abord, cette proposition de loi repose sur l'idée que les faits de corruption ont lieu exclusivement dans les pays les plus pauvres. Or cette idée est contredite par le rapport de l'OCDE sur la corruption transnationale

provenant de la vente de voitures de luxe, d'oeuvres d'art ou d'immeubles ayant servi à blanchir de l'argent détourné ou issues de la corruption soient reversées aux populations des pays où la corruption est- hélas ! -inscrite dans les moeurs et dans les habitudes. Pourtant, la proposition de loi qui nous est soumise ne répond pas encore à cette exigence morale. En effet, comme l'a souligné le rapporteur, la création d'un fonds au sein du budget général contrevient aux règles de la LOLF. Nous pouvons alors, mes chers collègues, regarder chez nos partenaires. L'affaire des biens mal acquis est un bon cas pratique : aux États-Unis, le, ou DoJ, a conclu un accord avec Teodorin Obiang Teodorin Obiang pour qu'il renonce à 30 millions de dollars d'avoirs qui seront reversés à des associations caritatives au bénéfice du peuple de Guinée équatoriale.

La Suisse, comme cela a été rappelé, est citée en exemple en matière de restitution des avoirs illicites : sur les trente dernières années, environ 2 milliards de dollars ont été restitués aux populations. L'évolution de la législation suisse est liée aux événements et présente un caractère d'opportunité.

Chaque fois, la Suisse s'engage dans un dialogue avec l'État concerné. Il n'y a donc aucune automaticité. Il faut le redire : l'automaticité de l'affectation des recettes pose question, puisque la moitié des affaires de corruption concerne les pays développés.

globale des missions de l'Agence. Il me semble que s'appuyer sur les ONG, comme le font la Suisse et les États-Unis, serait plus prometteur. Enfin, notre droit pénal mérite sans doute d'être revu, comme le suggèrent les auteurs de certains amendements. Malheureusement, la proposition de loi ne répond pas à ces questions juridiques.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je veux commencer par remercier Jean-Pierre Sueur de nous donner l'opportunité de discuter d'une question aussi importante que la corruption transnationale. Cette proposition de loi va dans le bon sens. Nous soutenons l'idée d'instaurer un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens détenus par des personnes étrangères, issus de la corruption transnationale. Nous soutenons l'idée de restituer ces sommes aux populations victimes. Oui, nous voulons être impitoyables avec celles et ceux qui accaparent les richesses de leurs peuples. Oui, la France doit être exemplaire. Nous pensons même qu'il est encore possible de renforcer la proposition

mes chers collègues, il est nécessaire d'éradiquer la corruption, cette « exploitation des gens sans défense » que condamnait l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun dans son recueil. S'engager contre ce S'engager contre ce phénomène est un impératif économique. Selon la Banque mondiale, chaque année, entre 20 et 40 milliards de dollars disparaissent dans les pays en voie de développement, soit l'équivalent de 20 % à 40 % de l'aide publique au développement.

L'OCDE, dans une étude de 2014, a souligné que ce sont majoritairement les directions d'entreprise et, dans 12 % des cas, directement les PDG, qui sont responsables des actes de corruption internationale. 11 % des personnages publics incriminés sont des présidents ou des présidentes, ou des membres de gouvernements ... Tous ces éléments revêtent un poids particulier pour notre pays. Oui, la France doit impérativement faire évoluer son arsenal juridique, car ses gouvernements successifs n'ont pas été exemplaires dans ce domaine- ne nous le cachons pas.

Dans ce contexte, cette proposition de loi va dans la bonne direction en prolongeant les acquis du droit international, et particulièrement les efforts de l'Organisation des Nations unies, sous les auspices de laquelle a été adoptée, en 2003, la convention dite de Mérida contre la corruption. Cependant, la nécessaire activation par l'État victime et le niveau parfois généralisé de corruption qui gangrène certains pays empêchent souvent l'application pleine et entière des principes de restitution et de et de partage direct avec les populations des avoirs issus de la corruption. De même, le partage n'est pas automatique : un accord est nécessaire avec l'État requérant. Dès lors, la restitution directe ou indirecte aux populations civiles fait trop souvent défaut. Le mécanisme contenu dans la proposition de loi pourrait résoudre ce problème.

Ensuite, nous souhaiterions que le mécanisme proposé intègre des perspectives de coopération avec les autres États mettant déjà en oeuvre ces procédures. Dans le même ordre d'idée, une évaluation annuelle de l'action du fonds devrait être réalisée et publiée, afin de nous permettre de suivre concrètement l'action des services de l'État. Les révélations sur les cas de corruption sont souvent le fruit du travail de journalistes, d'associations ou de lanceuses et lanceurs d'alerte. Ou des opposants ! Dès lors, nous revendiquons l'instauration d'une protection juridique dans le cadre des affaires de corruption transnationale. Enfin, nous pensons qu'une part importante des fonds récupérés, notamment ceux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une restitution, devrait participer directement au renforcement des systèmes fiscaux des pays en voie de développement.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur vise à traiter la question de la corruption transnationale, soit « l'accaparement de biens publics ou privés au profit d'une minorité d'oligarques d'une minorité d'oligarques qui bénéficient indûment d'un enrichissement illicite ». Les avoirs issus de la corruption transnationale procèdent pour l'essentiel de faits traduisant un manquement au devoir de probité devant guider les personnes dépositaires de l'autorité publique. L'équité exige donc d'affecter ces sommes détournées au profit des populations victimes de tels agissements, notamment au bénéfice des catégories les plus pauvres, privées des services de base- eau, électricité, santé ... -que leur État d'origine ne leur fournit La mise en oeuvre d'un tel principe est cependant loin d'être acquise. En l'état actuel de notre droit, rien ne permet en effet de garantir que les avoirs issus de la corruption transnationale soient restitués aux populations victimes ou, tout du moins, mis à leur bénéfice. Par l'effet de la décision de confiscation, ces fonds sont transférés au budget général de l'État en tant que recette non fiscale. Le Trésor public est donc le tout premier- voire l'ultime -bénéficiaire des avoirs issus de la grande corruption. C'est une situation difficilement acceptable qui constitue une double peine pour les populations victimes. La défaillance des gouvernements des États d'origine ne justifie en rien que ces avoirs, issus de la grande corruption, ne soient pas restitués aux peuples spoliés par leurs dirigeants malhonnêtes. Dès lors, il nous appartient d'adapter nos dispositifs législatifs, afin de garantir cette affectation. C'est une question de justice et d'honneur pour notre pays. Les juges français ont récemment marqué un pas décisif dans la lutte contre l'impunité de certains des anciens ou actuels dirigeants des pays concernés. Je pense notamment à la condamnation, en octobre 2017, du vice-président de Guinée équatoriale, Teodorin Obiang, à trois ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende, pour s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. L'ayant reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption, le tribunal a également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis, dont un somptueux hôtel particulier, situé avenue Foch, à Paris. Cette récente affaire met en évidence les enjeux majeurs qui demeurent autour de la restitution des avoirs. En effet, l'estimation du patrimoine confisqué s'élèverait à environ 150 millions d'euros, somme qui serait bien utile aux Équato-Guinéens Le coeur de cette proposition de loi permet d'aller plus loin en la matière en garantissant l'affectation des sommes confisquées non pas au budget général de l'État, mais bien à la restitution des avoirs illicites, conformément au principe plaidé par la France, voilà déjà quatorze ans, devant les Nations unies. Il existe une attente très forte de nombreuses organisations internationales et ONG, afin que la France garantisse l'affectation des sommes confisquées au bénéfice de l'amélioration des conditions de vie des populations, au renforcement de l'État de droit, ainsi qu'à la lutte contre la corruption dans le ou les pays concernés. Aujourd'hui, seule une minorité de pays, dont la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis, restitue aux populations des États d'origine les sommes confisquées dans le cadre d'affaires de corruption transnationale. Parmi ces pays, seule la Suisse s'est dotée d'une législation visant à restituer les valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger. Nos voisins helvètes ont ainsi pu restituer aux populations concernées près de deux milliards de dollars. Adopter la proposition de loi qui vous est soumise, mes chers collègues, constituerait une étape supplémentaire pour rendre justice aux populations victimes de la corruption. Notre collègue Antoine Lefèvre, rapporteur de ce texte, nous a indiqué partager les objectifs visés et a émis l'idée de faire transiter ces fonds par l'Agence française de développement.

Ce texte étant accueilli très favorablement par une très large majorité de nos collègues, nos discussions doivent permettre de lever les obstacles soulevés par la rédaction actuelle de cette proposition de loi.

grande complexité. En conclusion, à la veille du G7, sous présidence française, au mois d'août prochain, à Biarritz, l'adoption de cette proposition de loi par la Haute Assemblée enverrait un signal fort sur notre capacité à à traiter de ces délicates problématiques. Le groupe socialiste soutiendra ce texte et toute démarche qui permettrait de l'améliorer. La parole est

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, de l'avis de tous dans cet hémicycle, la corruption transnationale reste un fléau qui hypothèque l'avenir des populations des pays du Sud, au profit de quelques minorités confisquant les richesses. Notre devoir est de la combattre avec la plus grande détermination. Yvon Collin et le président Jean-Claude Requier se sont rendus, l'an dernier, au siège de la Banque mondiale, dans le cadre de leur mission de contrôle budgétaire des crédits de l'aide au développement. Ils y ont constaté non seulement l'absolue nécessité du système d'aide multilatéral, mais aussi sa trop grande complexité. Bien évidemment, les actions d'aide doivent être concentrées vers les pays les moins avancés. trop souvent, ce sont aussi ceux où le multilatéralisme comme la solidarité internationale sont aujourd'hui malmenés par les tensions géopolitiques et par diverses tentations de repli. La présente proposition de loi s'inscrit dans un contexte législatif et international où la lutte contre la corruption est, depuis plusieurs années, une priorité. Les États de l'OCDE ont adopté, en 1999, la convention de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales qui définit clairement la corruption transnationale comme l'accaparement de biens publics ou privés par une minorité de ressortissants d'États étrangers à des fins d'enrichissement illicite, dans l'intérêt d'acteurs, le plus souvent du Nord, visant à bénéficier d'accès indus à des marchés ou au commerce international. Par ailleurs, la convention des Nations unies contre la corruption, entrée en vigueur en 2005, a affirmé le principe de la restitution des avoirs acquis de façon illicite. illicite. En droit interne, la loi Warsmann, du 9 juillet 2010, a renforcé les conditions de saisie et de confiscation des profits illicites, en particulier en matière pénale, et a créé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Plus récemment, la loi Sapin II a introduit en France la convention judiciaire d'intérêt public qui permet de poursuivre plus efficacement les personnes morales soupçonnées de faits de corruption à l'étranger, comme cela se fait chez nombre de nos voisins. La proposition de notre collègue Jean-Pierre Sueur vise, quant à elle, les personnes physiques dites « politiquement exposées », c'est-à-dire des responsables étrangers mis en cause dans des affaires de biens mal acquis. Ce dossier a récemment connu des évolutions notables avec la condamnation du vice-président de Guinée équatoriale, en octobre 2017, à trois ans de prison et 30 millions d'euros d'amende pour détournement de fonds publics. Aujourd'hui, Rifaat al-Assad, oncle du président syrien Bachar al-Assad et ancien dignitaire du régime, pourrait également être inquiété pour des faits similaires. Il est vrai que les conditions de restitution des avoirs acquis illicitement continuent de poser d'importantes difficultés pratiques. S'il peut paraître injuste que l'État français saisisse purement et simplement des biens qui devraient, en toute logique, revenir aux États victimes de cette corruption, corruption, la persistance de la corruption dans ces États, voire l'absence de structure étatique digne de ce nom, rend hasardeuse toute entreprise concrète de restitution. À cet égard, j'émettrai quelques doutes sur l'efficacité de cette proposition de loi à atteindre réellement le but recherché, même si je souscris pleinement à son objectif. Le nouveau fonds serait ainsi chargé d'affecter les ressources récupérées « à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l'État de droit ainsi qu'à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions Mais les modalités précises de l'affectation sont renvoyées à un décret en Conseil d'État ... Pouvait-il en être autrement, compte tenu des contraintes strictes qui sont les nôtres en tant que parlementaires, du fait de l'article 40 de la Constitution et des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ?

Après ces remarques, et malgré quelques réserves, vous comprendrez, mes chers collègues, que les membres du groupe du RDSE voteront en faveur de cette proposition de loi. La parole

ils pourront comprendre et mesurer le rôle joué par les tiers et les fondations associées aux mécanismes de rétribution. Enfin, un dernier point ne devrait pas être négligé, celui des frais de procédure. Un rapport annuel permettrait d'éclairer la représentation nationale sur la fraction des sommes du fonds qui sont consacrées, aux enjeux de procédure. Le corollaire immédiat du principe de transparence est celui de l'efficacité. Le rapport annuel que je propose d'établir permettra de suivre l'évolution du fonds et, si besoin, d'adapter son fonctionnement. Au-delà même de l'action du fonds, il s'agira notamment de suivre les sommes affectées au budget général, qui sont impossibles à reverser.

En outre, en fonction de la mécanique budgétaire choisie, il ne semble pas nécessairement pertinent d'ajouter un tel rapport aux documents budgétaires existants. Enfin, il paraît nécessaire de préciser ce sur quoi porterait l'évaluation. Quel est

L'objet de ces amendements est de simplifier le régime des saisies et confiscations, d'améliorer l'action de l'Agrasc avant le jugement ou de faciliter l'indemnisation des parties civiles. Aussi pertinentes qu'elles puissent être, ces propositions nous éloignent de l'objectif premier de la présente proposition de loi, à savoir la restitution des biens mal acquis aux populations victimes. Compte tenu de ces éléments, la commission des finances a demandé le retrait de ces amendements, qui pourraient utilement trouver leur place dans le cadre d'une révision plus générale des dispositions pénales relatives aux saisies et confiscations et relèveraient à ce titre de la compétence de la commission des lois.

Merci